La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi

J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission d'enquête sur le contrôle, la régulation et l'évolution des concessions autoroutières a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle les explications de vote des groupes

collègues, à vous assurer que vous disposez bien de votre carte de vote et à vérifier que celle-ci fonctionne correctement en l'insérant dans votre terminal de vote.

Avant de passer au vote, je vais donner la parole à celles et ceux de nos collègues qui ont été inscrits pour expliquer leur vote. Le temps de parole imparti est de sept minutes

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, nous allons nous prononcer sur un texte qui va bouleverser les fondamentaux de notre société. En effet, qu'il s'agisse des liens parentaux et de la famille, du statut de l'embryon ou des manipulations génétiques, ce projet de loi suscite plus de questions qu'il n'apporte de réponses. assistée (PMA) sans père, il faut rappeler un principe évident : l'enfant n'est pas un droit que l'on exige et qu'il faudrait respecter à tout prix. Néanmoins, je précise qu'il s'agit non pas de priver les personnes d'avoir des enfants, mais de refuser la transformation de notre modèle de société pour des raisons compassionnelles. Par ailleurs, sous couvert d'égalité des droits, on oublie pourtant ceux de l'enfant, alors qu'il doit rester au centre des préoccupations. L'anonymat du donneur et l'absence de toute mention « né sous PMA » sur l'acte de naissance ne vont pas dans ce sens. Interdire à l'enfant d'avoir accès à son identité et à sa conception peut avoir de lourdes conséquences sur sa construction future. La PMA est fondée sur un principe d'égalité pour les femmes en couple ou célibataires, mais il faudrait aussi parler de l'égalité des droits pour les enfants. Connaître son père biologique et ses origines est un droit fondamental qu'on ne peut pas sciemment leur enlever par la loi. De plus, les obliger à attendre jusqu'à leur majorité pour connaître le donneur est une épée de Damoclès qu'on devrait leur épargner. Ce déni des droits de l'enfant a été encore aggravé par la dernière décision de la Cour de cassation, qui supprime de fait le contrôle sur les gestations pour autrui (GPA) réalisées à l'étranger. En éliminant la procédure d'adoption et en consacrant le parent d'intention, cette décision permet en réalité de contourner tout lien de filiation et donne la possibilité de le cacher complètement à l'enfant. Le Gouvernement est lui-même intervenu sur ce texte pour revenir à la loi actuelle et éviter les pires dérives des trafics d'enfants permis par cette décision. Concernant la GPA, nous savons tous que la PMA pour les couples de femmes induira nécessairement son autorisation au nom de l'égalité des droits. Dans ce cas, parlons aussi des droits des mères porteuses dans les pays en développement. La marchandisation du corps et l'exploitation de la pauvreté sont inacceptables. L'absence de contrôle dans ces pays affaiblit encore plus ces femmes face aux abus. Est-ce vraiment cela que nous voulons ? Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les dangers de ce texte, mais il faut conclure. Face à une série de mesures dont on ne maîtrise pas les conséquences et qui s'affranchissent des limites au nom du progrès, je voterai contre ce projet de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui amenés à nous prononcer sur un texte qui vient modifier sensiblement notre loi de bioéthique. Au terme de plusieurs heures de débat, nous avons abordé des sujets parfois troublants, souvent passionnants, toujours enrichissants. Je tiens à remercier les rapporteurs et le président de notre commission spéciale pour le travail accompli et la sérénité des débats. Nous avons participé à des discussions comme il y en a finalement assez peu dans cet hémicycle, appelant chacune et chacun d'entre nous à s'exprimer de manière transpartisane, à définir de nouvelles frontières pour l'avenir. Au sein de notre groupe, comme dans l'ensemble des autres groupes, nous ne nous sommes pas toujours accordés sur tous les sujets, tant ils sont sensibles : je pense particulièrement à la PMA ou encore au diagnostic préimplantatoire. J'ai moi-même évolué au cours des auditions, mais aussi du débat dans l'hémicycle. Sur d'autres dispositions, au contraire, un accord quasi unanime s'est dégagé. Je pense, bien sûr, aux évolutions sociétales que le texte initial prenait en compte pour mettre fin à une inégalité de traitement dans l'accès à la PMA entre couples hétérosexuels et couples de femmes. Comme je l'ai souligné lors de l'intervention générale, nous faisons partie de celles et ceux qui pensent que la PMA n'aurait pas dû figurer dans une loi de bioéthique ; mais le Gouvernement en a décidé autrement. Alors, nous avons bataillé pour que ce droit soit effectivement reconnu pour toutes, pour les couples de femmes et les femmes seules, et ce sans restriction, conformément au texte initial. C'est une avancée essentielle, qui reconnaît enfin

en séance, soit venue limiter le remboursement de l'acte aux seules demandes engagées sur la base d'un critère médical. Comment ne pas penser qu'il s'agit d'une concession aux anti-PMA, qui ont fait le siège devant le Sénat, nous inondant de méls prédisant la décadence de notre société ? Mes chers collègues, cette mesure ne peut souffrir de moitié d'égalité ! Si le texte reste en l'état, la situation actuelle ne se trouvera modifiée qu'à la marge : celles qui en ont les moyens

Drôle de conception d'une mesure censée rétablir une « inégalité » ... Comment ne pas nous indigner, également, de l'introduction d'une évaluation sociale et psychologique avant un recours à la PMA ? C'est totalement méconnaître le parcours des couples hétérosexuels, lesbiens ou de femmes seules candidats à la procréation médicalement assistée. C'est méconnaître le travail des équipes qui les suivent, les conseillent. Pourquoi une telle frilosité du Sénat, une attitude quelque peu punitive ? Malgré tous ces obstacles, la majorité du Sénat a heureusement voté en faveur de la PMA, ce qui pour nous était fondamental. Permettez-moi toutefois de souligner des reculs lors de l'examen de ce texte, qui nous ont fait nous interroger sur la finalité de notre vote au groupe CRCE. Ainsi, concernant le droit de la filiation : contre l'avis du Gouvernement, et de manière absolument conservatrice, la majorité est revenue sur le principe d'une reconnaissance conjointe anticipée, en privilégiant un processus d'adoption accéléré pour la « deuxième mère », ce qui ne va rien changer ou presque à l'existant. Pourtant, pour nous, le texte initial n'allait déjà pas assez loin. Dans les deux cas, on voit très bien les résistances à l'oeuvre, en ne mettant pas sur un pied d'égalité les parents hétérosexuels et les parents homosexuels. C'est aussi l'adoption qui a servi de base pour « laisser passer » l'article 4 sur l'interdiction de transcription totale à l'état civil des actes de naissance des enfants nés de GPA à l'étranger. J'en profite ici pour rappeler l'opposition de notre groupe à la GPA, qui, contrairement à la PMA, marchandise le corps des femmes. Cela dit, les enfants n'ont pas à être victimes de leur mode de conception et la loi doit permettre de leur apporter à tous une sécurité juridique. À ce propos, je ne peux que me réjouir, en tant que parlementaire communiste, que toutes les familles politiques aient dénoncé cette marchandisation des corps. Toutefois, il est édifiant de constater que cette unanimité ne s'appuie pas sur les mêmes approches idéologiques. Chez certains d'entre vous, mes chers collègues, il s'agit, comme chez les plus réactionnaires de nos concitoyens, de limiter la liberté de choix des femmes ! Preuve que le système patriarcal est toujours à l'oeuvre et qu'il faudra encore de nombreux combats pour en débarrasser la société. Toutes ces dispositions nous ont amenés à aborder l'accès aux origines. Au fil des débats, alors que nous étions plutôt favorables au texte de la commission spéciale proposant de laisser le libre choix aux donneurs de dévoiler leur identité aux 18 ans de l'enfant, nous avons finalement été convaincus par la version du Gouvernement ouvrant l'accès aux origines pour tous les enfants conçus avec tiers donneur. Il s'agit en effet d'abord d'une question d'égalité pour les enfants en question, sans parler de l'impact sur leur construction individuelle. Concernant la recherche, si certaines dispositions sont parfaitement autorisées à l'étranger, cela ne doit pas nous engager sur la piste du moins-disant éthique ; notre pays doit au contraire éclairer les autres nations avec son modèle bioéthique. Ainsi, l'utilisation des outils de modification ciblée du génome en recherche fondamentale ne doit pas être prise à la légère. Les dispositions proposées à l'article 17, que notre groupe a fait supprimer par voie d'amendement, mériteraient une discussion d'ampleur tant les questions soulevées posent éthiquement problème. Mais je pense personnellement que le Sénat a parfois été un peu trop timoré sur certaines dispositions ayant trait à la recherche, brandissant le risque d'eugénisme en confondant l'innovation avec les lignes rouges à ne pas franchir et la recherche sur un projet médical. Il en est ainsi du diagnostic préimplantatoire, à propos duquel, me semble-t-il, on a oublié le cadre étudié : l'infertilité des couples avec une réalité objective, à savoir que de nombreux embryons implantés n'iront pas jusqu'au bout. De ce point de vue, l'audition du professeur Frydman a été déterminante pour moi. En conclusion, ce texte porte en lui toute une vision de la société et du sens que l'on veut donner à l'évolution de l'espèce humaine sur notre planète. La navette va se poursuivre et elle va contribuer, pour une fois, de mon point de vue, à corriger bon nombre des reculs que je viens rapidement de dénoncer. Nous voterons donc en faveur de ce projet de loi, en restant très vigilants. À nous de continuer à réfléchir, sans, sur le monde de demain, tel que nous contribuons à le dessiner, pour espérer le rendre meilleur, en nous affranchissant en nous affranchissant des maux qui caractérisent notre société moderne et capitaliste. Mes chers collègues, il s'agit au fond de prendre de la hauteur sur ces enjeux scientifiques et sociétaux, pour avoir une approche qui ne soit ni déshumanisante ni discriminante. C'est ainsi que nous serons une société éthique.

qui surgissent de la science. Nous révisons ces lois régulièrement, à un rythme qui d'ailleurs s'accélère pour s'ajuster aux avancées de la médecine, de l'intelligence artificielle et de la science en général. Le groupe Les Indépendants tient à saluer le travail de la commission spéciale, de ses rapporteurs et de son président. Nous souhaitons aussi féliciter l'ensemble de nos collègues pour la qualité des échanges que nous avons eus : nos positions étaient diverses, mais nous avons su nous écouter les uns les autres et maintenir le débat à la hauteur des enjeux. Nous avons ainsi su garder au coeur de nos débats la bienfaisance, que l'on retrouve dans l'injonction d'Hippocrate : « D'abord, ne pas nuire. » Nous avons aussi été attentifs au respect de la dignité de la personne humaine, comme le prévoyaient déjà les lois de 1994.

a été voté et a été aussi amendé. La PMA est donc autorisée pour les couples de femmes et les femmes seules. Plusieurs de ses modalités ont été modifiées. Le financement de cet acte, d'abord : notre assemblée a souhaité limiter le remboursement de la PMA par la sécurité sociale aux seuls couples hétérosexuels infertiles. Avant la réalisation de cette PMA, le Sénat a aussi souhaité la mise en place d'une évaluation psychologique. Si le Comité consultatif national d'éthique s'est montré favorable à cette loi, l'Académie nationale de médecine et le Conseil de l'ordre se sont interrogés sur les effets de l'absence de père sur l'enfant, sans s'opposer néanmoins à la PMA. Quant à la précarité d'une femme seule qui y recourrait, il faut indiquer que celle-ci ne sera pas toujours acceptée par l'équipe médicale. De plus, il s'agit une monoparentalité choisie et non subie. Le Sénat a également exclu les PMA. À titre personnel, je suis favorable à cette rédaction de l'article 1. Nos débats ont été l'occasion d'entériner le fait qu'il n'existe pas de droit à l'enfant. Le Sénat a aussi supprimé la possibilité de réaliser un diagnostic préimplantatoire.

Le maintien de l'interdiction de tous les tests génétiques a été décidé par notre assemblée. Je pense qu'il aurait mieux valu les encadrer, car ils sont de toute façon disponibles sur internet. À l'article 2, le Sénat a supprimé l'autoconservation des gamètes pour des raisons de pression sociale. Personnellement, je ne pensais pas que les comportements de certains employeurs puissent être aussi violents. Sur une autre mesure phare,

qui en fait la demande pourra connaître l'identité du donneur, sous réserve que ce dernier y consente. Dans le cas d'un couple de femmes, la filiation reconnaissance conjointe devant un notaire a été remplacée par la voie de l'adoption. J'ai voté cet amendement. La PMA et le don de gamètes sont deux sujets ayant un fort retentissement dans notre société. Le projet de loi comporte d'autres dispositions qui ne sont en rien secondaires. C'est le cas des dispositions encadrant la recherche sur les embryons, les cellules souches humaines et les cellules pluripotentes humaines. a supprimé les embryons chimériques animal-homme et homme-animal, et le Sénat l'a suivie sur ce point. La possibilité d'introduire des cellules pluripotentes dans l'animal a été rejetée. Le Sénat a fait le choix d'autoriser, à titre dérogatoire, les recherches sur les embryons jusqu'à leur vingt et unième jour de développement. Il faut rappeler que les recherches se font sur des embryons non implantables, avec l'accord du couple. Cette recherche vise à étudier la gastrulation et, ainsi, à comprendre la différenciation des cellules à ce stade, ce qui est très important pour la recherche et les applications médicales. Au-delà des problématiques liées à la recherche, le texte comporte également des dispositions qui touchent les Français dans leur quotidien. Je pense notamment aux dons d'organes, de cellules hématopoïétiques et de sang, qui sont facilités par l'article 5. Notre assemblée a aussi confirmé la suppression du délai de réflexion du couple en cas d'interruption médicale de grossesse. Si ce projet de loi n'a jamais comporté de disposition autorisant la GPA, le Sénat a fait le choix d'insérer un nouvel article afin d'interdire la transcription d'actes étrangers mentionnant un ou des parents d'intention dans les registres de l'état civil. J'ai voté cet amendement. ne peut pas être résumé à ces mesures et bien d'autres sujets y ont été abordés. Nous avons vu au cours des débats que toutes ces questions dépassent les clivages politiques actuels appliquer la loi de bioéthique tout en permettant des avancées sociétales et en matière de recherche médicale. Chacun votera conformément à ses valeurs, à ses idées, mais aussi à ses croyances. À titre personnel, je suis globalement favorable aux évolutions apportées par ce projet de loi, même si je regrette certaines suppressions. J'ai bien conscience de ne pas représenter la diversité des opinions de mon groupe.

de tous leurs interlocuteurs, ils ont su faire preuve d'un sens de l'écoute particulièrement remarquable. Grâce à eux, le Sénat a su ouvrir à un large spectre les consultations menées pour le plus grand bénéfice du débat démocratique. Permettez-moi également de me faire l'interprète de nombre de mes collègues en soulignant, madame la ministre, combien pouvoir débattre d'un sujet majeur comme celui-ci sans pâtir des inconvénients inhérents à la procédure accélérée est appréciable. Voilà pour ce qui est de la forme. Quant au fond, la commission spéciale a donc adopté ce texte en y apportant de substantielles modifications, puisqu'elle l'a enrichi de 137 amendements. Le texte final, aux conséquences considérables sur un plan tant médical que « sociétal », a, pour l'essentiel, lors de l'examen en séance publique : adopté, avec modification, l'extension de l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules ; rejeté l'autorisation d'autoconservation de gamètes sans raison médicale ; adopté, avec modification, l'accès aux origines modifié l'établissement de la filiation d'un enfant issu d'une AMP par un couple de femmes ; donné une portée pleine et entière à l'interdiction de la gestation pour autrui ; rétabli l'interdiction de la création d'embryons transgéniques transgéniques ; et soutenu l'ouverture de la possibilité de tests génétiques en première intention dans le cadre du dépistage néonatal. Permettez-moi d'ajouter que, lors des débats, en confirmant le texte de la commission spéciale à l'article 3 concernant l'accès aux origines des personnes nées d'un tiers donneur, nous avons trouvé un point d'équilibre facilitant l'accès aux origines tout en protégeant l'identité des donneurs. L'article 4, sur la filiation d'un enfant issu d'une AMP par un couple de femmes, quant à lui, été entièrement récrit. Il interdit désormais l'établissement de deux filiations maternelles concernant un même enfant tout en modifiant les conditions requises pour l'adoption, afin d'en permettre la réalisation par la mère d'intention. Sur ce point précis, madame la ministre, ce dispositif permet, comme dans le texte que vous proposiez, d'apporter une réponse au nouveau fait social autorisé par l'article 1. certains au groupe Union Centriste s'interrogent sur la capacité de ce dispositif à répondre à la demande sociétale qui est exprimée par les couples de femmes. Enfin, l'article 4 a ouvert la discussion sur la GPA. Le Gouvernement, opposé à la suppression de cet article, a montré qu'il partageait notre préoccupation. Cependant, plusieurs de mes collègues ne jugent pas le texte satisfaisant dans la mesure où il traite simplement de mesures juridiques et administratives relatives à l'état civil, ce qui n'est donc pas susceptible d'empêcher les couples d'y avoir recours. Pour poursuivre, c'est avec l'avis favorable, sinon le soutien du Gouvernement, que le Sénat a supprimé l'ouverture des tests génétiques pour tous, les tests génétiques à visée généalogique ou encore les diagnostics préimplantatoires avec recherche d'aneuploïdies. L'adoption de l'article 14 permet à la recherche sur les cellules souches embryonnaires de répondre à un régime de déclaration et porte, par ailleurs, la durée possible de la recherche sur l'embryon de sept à quatorze jours et, par dérogation, à vingt En outre, la suppression de l'article 17, qui posait le principe de l'interdiction de création d'embryons chimériques humains tout en ouvrant la création de chimères par adjonction de cellules souches pluripotentes humaines sous certaines conditions, a été supprimée. les dispositions de cet article devant être considérées au regard de celles de l'article 4, qui n'ont pas été modifiées en conséquence, certains, parmi mes collègues, s'inquiètent de l'imprécision potentielle du cadre juridique relatif à la recherche sur les chimères tel qu'il ressort de nos travaux. C'est ainsi qu'à l'issue de nos travaux en première lecture, à l'article 1, nous avons collectivement choisi de permettre l'extension de l'AMP tout en en précisant les conditions et interdit le double don de gamètes. Paradoxalement, alors que l'AMP n'a toujours été autorisée qu'en cas d'infertilité ou de risque médical, l'interdiction du double don de gamètes cumulée à la suppression de ce critère aboutit au fait que la femme seule fertile pourra recourir à l'AMP, tandis que la femme stérile ne le pourra pas. C'est le choix que nous avons fait majoritairement, mais pas unanimement. De la même manière, la prise en charge par l'assurance maladie n'est désormais possible que dans les cas d'AMP fondées sur des indications médicales. Pour ce qui est de l'article 2, en supprimant l'autoconservation des gamètes sans raison médicale, nous avons voulu protéger les femmes d'éventuelles pressions de leurs employeurs. Enfin, le diagnostic préimplantatoire avec type HLA, ouvert depuis 2004, a été confirmé. Ainsi, comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, les discussions ont été sérieuses et approfondies, et les sénateurs du groupe Union demeurent partagés sur le texte issu de cette première lecture. Pour ma part, et les amendements que j'ai déposés en témoignent, je suis et reste un opposant à la PMA, notamment parce qu'elle est l'antichambre de la GPA. Tout à fait ! Soyez assurés, mes chers collègues, que je ne suis en rien réfractaire à la marche

Nos choix refléteront nécessairement un certain état de la science, des mentalités et de l'éthique. Ils résulteront de la confrontation entre le possible et le souhaitable, entre des parcours individuels parfois douloureux et des conséquences collectives. C'est au Parlement

car votre conception de la filiation n'est pas et ne sera jamais la mienne, tant elle va à l'encontre des principes fondamentaux qui s'attachent à la dignité humaine. Les enfants naissent d'êtres humains et doivent rester des êtres humains, avec leur beauté et leurs imperfections ! La parole

Ce vote ne sera pas unanime. Vous n'en serez pas surpris. Ce vote ne sera pas unanime, peut-être parce que certains- ce n'est pas mon cas -estiment qu'on a, à tort, associé, dans ce projet, une décision sociétale, qui est l'extension de l'assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes,

nous avons rappelé que la sécurité sociale a pour vocation de rembourser non pas des actes médicaux, mais bien des actes en lien avec les risques et les conséquences d'une maladie. Deuxièmement, nous avons rappelé que l'égalité des familles tient plus à l'égalité des droits et des obligations entre les parents et les enfants qu'à l'identité des modes de filiation. la raison pour laquelle, dans les couples de femmes, les mères auront les mêmes droits et obligations à l'égard des enfants, mais ne bénéficieront pas du même mode d'établissement de leur filiation : celle qui a accouché sera la mère, quand l'autre deviendra mère en adoptant l'enfant. Sur ce point, nous avons donc fait preuve de cohérence juridique. Enfin, nous avons rappelé que, pour que l'interdiction de la gestation pour autrui qui existe en France soit effective, il ne fallait pas que l'on puisse transcrire l'intégralité des actes d'état civil établis à l'étranger à l'issue de GPA qui y sont réalisées. La deuxième ligne directrice que nous pouvons retrouver dans ce projet est constituée par les choix éthiques que nous avons arrêtés, qui établissent les limites que la condition humaine doit fixer à la science. Ainsi, nous avons supprimé le dépistage préimplantatoire, sur les embryons, des anomalies chromosomiques. Nous avons maintenu les limites du diagnostic préconceptionnel. Nous avons interdit les modifications génétiques ainsi que l'introduction des cellules humaines dans un embryon animal- autrement dit, nous avons interdit les embryons transgéniques et les embryons chimériques.

C'est la raison pour laquelle les débats ont été importants, comme l'ont dit Muriel Jourda ou encore Laurence Cohen. Ils ont été intenses. Ils ont fait état de notre diversité et des interrogations de chacun. Dans chaque groupe existe, bien évidemment,

souvent citée- c'est l'une des rares à évoquer ce point -, insiste, en son article 28, sur la nécessité du débat public : « Les parties à la présente convention veillent à ce que les questions fondamentales posées par les développements de la biologie et de la médecine fassent l'objet d'un débat public approprié à la lumière, en particulier, des implications médicales, sociales, économiques, éthiques et juridiques pertinentes, et que leurs possibles applications fassent l'objet de consultations appropriées. » C'est la raison pour laquelle

devait être « une loi de confiance dans l'individu sur les grandes avancées des sciences plutôt qu'une loi d'interdiction ». Ce texte, mes chers collègues, ne répond sans doute pas à ce voeu. Ainsi, le titre I ne

Fort heureusement, les amendements que nous avons proposés en commission ont rejoint les propositions des rapporteurs Olivier Henno, Corinne Imbert et Bernard Jomier,

du CCNE. Franchement, votre titre III- « Appuyer la diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques » -est complètement en deçà des réalités. En fait, le Gouvernement a souhaité limiter considérablement cette diffusion. Restent quelques petites lueurs d'espoir dans le titre IV, « Soutenir une recherche libre et responsable au service de la santé humaine ». Mais que fait-on de procès aux chercheurs !

Sur ces sujets qui touchent à l'intime, je tiens à souligner la qualité des débats qui se sont tenus ces deux dernières semaines, avec l'éclairage indispensable de nos quatre rapporteurs, dont je salue le travail.

Cette troisième grande révision des lois de bioéthique a été l'occasion pour nous d'évoquer des sujets aussi sensibles que la naissance, la mort, la maladie, le désir d'enfant, l'intérêt de l'enfant et, ainsi, des barrières éthiques que nous souhaitons poser aux progrès de la science. Quand je dis « nous », je parle de la société tout entière, mais aussi des sénateurs qui composent cette assemblée et qui s'efforcent, avec conviction, de la représenter. Comme on l'a vu tout au long de ses débats, il n'est pas aisé, pour un parlementaire, de trancher sur des sujets aussi sensibles. Il y a eu, chez certains, une forme d'appréhension légitime à l'approche de l'examen Mais c'est le choix qu'a fait la France de confier aux représentants du peuple la responsabilité d'ériger des lignes rouges à ce que la science peut faire, considérant que l'élection démocratique nous octroie cette légitimité, qui ne vaut en aucun cas mandat impératif. C'est aussi au travers de la diversité de nos valeurs, de notre propre histoire et de celle de nos familles que nous sommes en capacité d'énoncer l'interdit. C'est portés par cette complexité que nous nous sommes astreints à légiférer en gardant toujours à l'esprit l'intérêt général, ce que nous comprenons de la société et ce que celle-ci souhaite pour son avenir.

Ma propre éthique m'a poussée à défendre, tout au long des débats, la capacité des femmes à décider de ce qui est bon pour elles et pour leur enfant à naître, à respecter leur désir de parentalité et leur résistance aux différentes pressions sociales qui s'exercent. Aussi, j'ai deux grands regrets à l'issue de cette première lecture. Premièrement, pour que la procréation médicalement assistée soit un droit réel pour toutes les femmes, il est indispensable que le remboursement ne soit pas restreint aux seules demandes fondées sur une pathologie médicalement prouvée d'une part, parce que l'on maintiendrait alors une rupture d'égalité entre les femmes qui peuvent payer et celles qui ne le peuvent pas ; d'autre part, parce que la cause de l'infertilité n'est pas toujours médicalement prouvée, y compris pour les couples hétérosexuels. s'agissant de la conservation des ovocytes, le vote s'est malheureusement cristallisé autour de la possibilité- ou de l'impossibilité -de réaliser cette procédure dans des établissements privés privés à but lucratif. Le RDSE a voté en majorité contre l'article 2, par rejet non pas de l'autoconservation ovocytaire, à laquelle il était favorable, mais d'une procédure qui, si elle était effectuée dans des établissements à but lucratif, ferait craindre à la majorité d'entre nous une forme de marchandisation qu'elle refuse. Le débat, quant à lui, s'est concentré sur les pressions sociales subies par les femmes, pressions qui s'accentueraient en cas de généralisation de l'autoconservation de gamètes. Il est peut-être vrai que les femmes subissent des pressions sociales, tantôt pour fonder une famille, tantôt pour privilégier leur carrière. Il est salutaire d'en débattre, mais pas de les brandir comme un argument suffisant à justifier l'incapacité des femmes à décider pour elles-mêmes. Aussi, j'espère que la deuxième lecture nous permettra de nous entendre sur une rédaction plus ouverte sur l'autoconservation des ovocytes sans critère médical. Trois autres sujets méritent un commentaire en lien avec la PMA, notamment la fécondation. Si les débats sur la PMA ont été empreints de beaucoup de respect et de dignité, je suis favorable, comme je l'ai exprimé, à son autorisation et ne peux donc pas me réjouir du vote, très serré, qui a conduit à son rejet. Il en est de même pour le double don de gamètes, qui pourrait offrir une réponse aux couples doublement infertiles, et pour le diagnostic préimplantatoire pour la recherche d'aneuploïdies, lequel permettrait aux femmes ayant subi de nombreux échecs de limiter les risques de fausses couches lors de l'implantation de nouveaux embryons. J'en viens maintenant aux questions de filiation. Si je suis farouchement opposée à l'article 4, introduit en commission, qui pénalise l'enfant né d'une GPA à l'étranger, en interdisant la transcription de son acte de naissance en droit français, je regrette également le choix fait par la majorité sénatoriale concernant l'établissement de la filiation dans le cas des PMA réalisées pour les couples de femmes. La rédaction initiale de l'article 4 semblait tout à fait satisfaisante, en permettant la double filiation maternelle par déclaration anticipée de volonté, tandis que la filiation par adoption pour la mère d'intention ne me semble pas aller dans le sens du progrès. Pour terminer, je veux saluer l'interdiction, votée en séance publique, des tests génétiques à visée commerciale. Des doutes demeurent, me semble-t-il, sur la fiabilité et la confidentialité de ces tests et des données récoltées. Après les débats, qui ont été riches et argumentés, je reste convaincue que le recueil d'informations génétiques doit rester circonscrit au milieu médical. En résumé, comme l'ont dit

Si mon propos liminaire faisait l'éloge de nos débats et ma revue des articles mentionnait de nombreux désaccords avec la majorité sénatoriale, ma conclusion fait la synthèse du rôle qui a été le nôtre ces deux dernières semaines : nous avons dû faire des choix, prendre des décisions qui impacteront la vie intime de nombreux Français. Pour eux, le groupe RDSE ne peut se résoudre à rendre une copie blanche. Nous avons débattu en bonne intelligence. Les conditions ont été réunies pour l'examen de sujets aussi sensibles que complexes. Nous ne pouvons donc nier ce débat qui a eu lieu et les avancées notables qu'il a fait émerger, malgré nos nombreux désaccords. C'est pourquoi le groupe RDSE votera en majorité pour l'adoption de ce texte. Et, puisque l'occasion nous est donnée- une fois n'est pas coutume -d'examiner un projet de loi en procédure normale, et non en procédure accélérée, nous profiterons de la deuxième lecture pour tenter de vous convaincre. La parole

Comme dans chaque groupe, des convictions personnelles divergentes se sont exprimées, tant les mesures contenues dans ce texte se situent à la croisée de chemins philosophiques, scientifiques, médicaux et sociétaux. Les nombreuses mises au point au sujet de votes en témoignent. De ce point de vue, notre groupe n'a pas fait exception. Au cours de l'examen du projet de loi, nous avons abordé certains sujets avec des convictions fortes, sans toujours réussir à les faire partager. Je pense bien évidemment à l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation à toutes les femmes. Je reste, pour ma part, convaincu de la justesse de cette mesure. Les réticences des uns et des autres sont non pas éthiques, mais culturelles, voire cultuelles. Je suis, à ce titre, déçu- oui, déçu ! -que le Sénat ait ouvert un droit nouveau pour aussitôt en restreindre l'accès, en réintroduisant le critère pathologique et en excluant, ce faisant, les femmes seules ou les couples lesbiens du remboursement par l'assurance maladie. Permettez-moi de rappeler qu'actuellement 15 % des couples hétérosexuels qui recourent à l'AMP ne présentent aucune infertilité médicalement constatée. Devra-t-on les exclure du recours à cette technique ? Qu'en sera-t-il également des couples qui, après avoir recouru à une AMP, ont un enfant naturellement ? Avec le système que vous avez mis en place, seront-ils contraints de rembourser la sécurité sociale ? Qu'est-ce qui empêchera les femmes de continuer à se rendre à l'étranger et de se faire rembourser en France, comme c'est déjà le cas ? Vous voyez bien que cette exclusion ne tient pas la démonstration et qu'elle cherche à induire une rupture d'égalité d'accès au droit, en distinguant celles qui auront les moyens des autres ! Je le réaffirme : l'extension de l'AMP à toutes les femmes n'opérera pas de glissement irréversible vers la gestation pour autrui. L'Espagne et la Norvège n'ont pas autorisé la GPA. En revanche, l'Estonie et la Lituanie, qui l'ont permise, refusent l'AMP aux couples de femmes. À l'occasion de ces débats, nous avons tous, à quelques rares exceptions près, pu rappeler notre opposition farouche à la GPA, laquelle est laquelle est interdite dans notre pays à tout le monde, ainsi que notre préoccupation pour le sort des enfants qui en sont issus. Une telle précision dans ce débat m'est apparue inutile, tout comme celle qui vise à rappeler que nul n'a de droit à l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant a d'ores et déjà valeur constitutionnelle et supraconstitutionnelle. Où est cet intérêt lorsque l'on s'oppose à la transcription totale dans les actes d'état civil des actes de naissance de ceux qui sont nés à l'étranger à la suite d'une GPA ? S'agissant de la levée de l'anonymat du donneur ou de la donneuse de gamètes, que l'on oublie trop souvent, à l'égard de l'enfant issu d'un don, il me paraît cruel et inégalitaire de laisser ce dernier dans l'incertitude jusqu'à sa majorité. Mettre fin à la tourmente à laquelle peut- je dis bien « peut » -exposer la quête de ses origines, c'est précisément ce que le texte cherchait à faire. Enfin, je continue de croire que l'autoconservation des gamètes n'incitera pas les femmes à reporter leur grossesse. Elle leur donnera, au contraire, une chance supplémentaire de préserver leur fertilité jusqu'à ce qu'elles rencontrent un partenaire sérieux.

Cessons de traiter les femmes comme de petites choses fragiles qui auraient besoin d'être protégées de tous, y compris d'elles-mêmes, et laissons-les disposer enfin de leur corps Nous regrettons également que le Sénat ait rejeté la possibilité d'insérer des cellules souches pluripotentes induites humaines, les « cellules iPS », dans un embryon animal, malgré un encadrement très strict. Cette technique aurait permis à la recherche de faire un véritable bond. Cela traduit Cela traduit une véritable défiance vis-à-vis du monde scientifique, jugé au mieux désinvolte, au pire dénué de discernement éthique. Je ne m'y associe évidemment pas., de doutes que nous avons examiné d'autres sujets. Nous avons même, parfois, changé de conviction au cours de nos discussions. Je pense aux débats de très grande qualité qui ont eu lieu, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, autour de l'AMP ou encore ou encore sur l'expérimentation de l'accès aux examens génétiques. Ils ont, je le crois, fait honneur à la représentation nationale. Pour d'autres mesures, les solutions trouvées ne nous satisfont pas encore. C'est le cas du mode de filiation retenu pour les enfants ayant deux mères. Nous aurions souhaité placer tous les parents dans une situation d'égalité. Le Gouvernement n'ayant pas déclaré l'urgence sur ce texte, la navette nous permettra de poursuivre nos réflexions pour, je l'espère, y parvenir. Je pense sincèrement que ce texte, qui est l'aboutissement d'un long travail de consultations mené par le Gouvernement pour mettre à jour la législation en matière de bioéthique, contenait initialement des avancées scientifiques et sociétales majeures, dans le respect de ce qui fonde notre éthique. Madame la ministre, vous l'avez rappelé, il n'y a pas, d'un côté, les garants de l'ordre moral et, de l'autre, ceux qui, au nom d'une liberté et d'une égalité débridées, conduiraient à sa perte. Mais nous ne pouvons nous résoudre à voter contre une avancée des droits, une avancée sociétale telle que l'extension de l'AMP pour toutes. Nous sommes attendus sur cette promesse présidentielle : au-delà de ces murs, de nombreuses femmes nous regardent

Ces débats nous ont montré que le patriarcat et le paternalisme avaient encore de beaux jours devant eux. En définitive, puisqu'il est hors de question de laisser la place au doute, les symboles tels que l'AMP étant encore plus importants que les nombreux reculs votés au Sénat, le groupe La République En Marche, dans sa majorité, votera en faveur de ce projet de loi.

dans le terminal. Je vous rappelle que, si vous disposez d'une délégation de vote, le nom du sénateur pour lequel vous devez voter s'affiche automatiquement sur le terminal au-dessous de votre nom. Vous pouvez alors voter pour vous et pour le délégant en sélectionnant le nom correspondant, puis en choisissant une position de vote. Si vous avez donné une délégation et que vous êtes finalement présent, vous pouvez voter directement en insérant votre carte dans votre terminal de vote. La position de vote alors exprimée primera sur un vote exprimé par délégation.

à constater le résultat du scrutin.

madame la ministre Monsieur le président, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs,

la dimension tout à fait singulière de ce texte et les conséquences concrètes qu'il emportera, demain, sur la vie de nos concitoyens. C'est la grandeur du Parlement que d'assumer un certain nombre de changements que la science rend possibles et que la société appelle.

dernières semaines, nous avons cheminé ensemble sur la ligne de crête qui sépare le possible du souhaitable. Je le répète, c'est aux représentants de la Nation de discerner et d'établir la frontière entre ces deux mondes.

je me réjouis que cette assemblée reconnaisse la famille dans ce qu'elle a de divers, de pluriel et de riche. J'ai une pensée toute particulière pour ces familles dont le projet de vie qu'elles construiront sera reconnu, bien au-delà de l'affection de leurs proches, par les lois de la République et au travers des droits et des devoirs que ces lois donnent à chacun. Ces familles nous regardent peut-être ; je sais qu'elles nous attendent. Voilà deux semaines, lors de la discussion générale, j'avais indiqué qu'aucune des mesures de ce projet de loi ne devait mettre en tension le moindre principe éthique fondamental. C'est à ce titre que j'ai proposé la suppression des dispositions relatives à la génétique introduites par la commission spéciale. Je reste convaincue que le temps est encore à la recherche, pour mieux comprendre l'impact des différentes mutations génétiques et leurs conséquences non seulement en termes de prévention et de soins, Les nouveaux droits qui seront ouverts par le texte ne doivent être contraires à aucun principe bioéthique et ne peuvent s'exercer que dans un cadre protecteur. les modifications que vous aviez apportées à l'article 2 et l'ouverture de l'autoconservation aux centres privés ne garantissaient plus ce cadre protecteur. Je pense sincèrement qu'il était préférable de ne pas adopter cet article ainsi modifié, ce que vous avez fait.

Nous souhaitons reconnaître un projet parental porté par deux femmes. Il n'y a aucune raison d'imposer à l'une d'elles de passer par l'adoption. Le système que nous proposons permet de sécuriser l'établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant et de ses deux mères.

la conformité de la transcription de l'acte de naissance de l'enfant s'apprécie au regard des critères de la loi française. Cette solution, plus générale que celle qui a été adoptée, englobe un plus grand nombre de cas. Il est hors de question, je le rappelle solennellement, de légaliser la GPA. Nous y sommes farouchement opposés. L'enjeu est ici de trouver un équilibre entre l'effectivité de l'interdiction de la GPA en France et la nécessaire reconnaissance d'un état civil sécurisé pour des enfants qui ont le droit de voir leur filiation établie et de vivre une vie familiale normale. Frédérique Vidal et moi-même avons décidé de relever d'emblée les points susceptibles de déséquilibrer le texte ou de l'entraîner dans une direction qui ne nous semble pas opportune. Les recherches sur l'embryon humain telles que nous les défendons doivent avoir pour seul objectif d'enrichir nos connaissances de la biologie de l'homme et d'améliorer la santé. J'observe que les articles qui concernent la partie recherche ont été profondément modifiés. Je ne doute pas que le débat sera encore dense lors des prochaines lectures. les sénateurs, un certain nombre de sujets seront approfondis lors des prochaines navettes parlementaires, mais je voudrais saluer une nouvelle fois la qualité, la sincérité et la richesse de nos débats, malgré les divergences

sujets sont majeurs pour nous. Nous ne sommes pas que la chambre des collectivités territoriales, nous sommes la chambre de la société française et des citoyens ! Mes chers

La séance est reprise. Mes chers collègues, par lettre en date du 3 février, le Gouvernement demande l'inscription de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à modifier les modalités du congé de deuil pour le décès d'un enfant à l'ordre du jour du mardi 3 mars après-midi, après le vote solennel sur le projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée. Acte est donné de cette demande. Le délai limite de dépôt des amendements de séance pourrait être fixé au lundi 2 mars, à midi, et le temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale serait d'une heure. Y a-t-il des observations ?

président du groupe Les Républicains, demande le retrait de l'ordre du jour du jeudi 20 février du débat, inscrit à la demande de son groupe, sur le programme de travail de la Commission européenne et sur les perspectives de l'action européenne d'ici 2024 et son remplacement par un débat sur l'action du Gouvernement en faveur de l'agriculture. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi modifiant les lois du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution

celui d'accéder à un service minimum garanti, c'est-à-dire effectif, dans les transports publics. Il s'agit de tenir compte de l'exaspération de tant de nos compatriotes qui se retrouvent

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'épisode de grève d'une durée sans précédent dont notre pays sort à peine est venu rappeler que l'absence de certains services publics, notamment en matière de transports,

La paralysie des transports publics a entraîné des difficultés parfois considérables pour nos concitoyens habitant loin de leur lieu de travail. Ceux qui en ont les moyens ont dû assumer des frais d'hébergement ou de garde d'enfant. Mais les personnes les plus affectées ont été les plus fragiles, celles qui ne pouvaient pas se passer d'aller travailler, qui n'ont pas pu se permettre de prendre des jours de congé ou qui n'ont pas d'autre solution de transport que le train, le bus, le métro. Ce sont d'abord à ces personnes que nous devons penser lorsque nous légiférons Cette situation s'est traduite par un regain du recours aux transports individuels, à l'heure où la promotion des transports collectifs apparaît comme une réponse essentielle aux enjeux environnementaux. On peut craindre que beaucoup, parmi ceux qui se sont reportés sur la voiture individuelle, gardent désormais ce mode de transport et ne reviennent pas aux transports en commun. Si la situation s'est aujourd'hui nettement améliorée, cette expérience encore bien présente dans nos mémoires doit nous pousser à nous interroger sur les moyens de garantir la continuité du service public et, plus largement, d'assurer la couverture des besoins essentiels de la population. de grève est un droit constitutionnel, il n'est pas un droit absolu, et il n'est pas supérieur aux autres droits et principes de valeur constitutionnelle. C'est ce qu'a jugé avec constance le Conseil constitutionnel, estimant que le droit de grève

Le législateur a ainsi pu prévoir des aménagements du droit de grève. Dans le secteur public, il a prévu une obligation de préavis et a même privé certaines catégories d'agents du droit de grève. le même sens, la loi prévoit d'ores et déjà la possibilité de requérir des personnels grévistes dans certains cas précis : cette possibilité est ouverte au Gouvernement, en vue de préserver la sécurité nationale, et au préfet, lorsqu'une atteinte à l'ordre public l'exige. Ces possibilités de réquisition concernent tant des agents publics que des salariés d'entreprises privées, et dépassent même le seul cas du service public. Dans le secteur des transports publics, la loi du 21 août 2007 a prévu un encadrement spécifique. Ainsi, le dépôt d'un préavis de grève doit être précédé du déclenchement d'une procédure d'alarme sociale, et les salariés souhaitant se mettre en grève sont tenus de le déclarer à leur employeur au moins quarante-huit heures à l'avance. Ces dispositions ont permis d'améliorer le dialogue social et de donner aux usagers une information fiable sur le service assuré. Pour autant, la loi de 2007 rencontre ses limites lorsqu'un conflit trouve son origine dans des décisions sur lesquelles l'employeur n'a pas de prise. En outre, si elle définit différents niveaux de service en fonction de la perturbation, elle ne permet pas d'assurer un service minimal à même de couvrir les besoins essentiels de la population en cas de grève très suivie.

Il s'agit non plus de partir du service qui peut être assuré compte tenu du nombre de grévistes, mais bien de partir des besoins essentiels de la population et de prévoir les moyens d'assurer la couverture de ces besoins. Le texte crée un droit pour les usagers à un service minimum de transport en cas de grève et ne limite le droit de grève que dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir ce service La commission des affaires sociales, partageant largement cet objectif, a adopté ce texte en lui apportant plusieurs modifications destinées à sécuriser ses dispositions. L'article 3 de la proposition de loi, qui en constitue le coeur, fixait le niveau minimal de service à un tiers du service normal, concentré aux heures de pointe, ce niveau pouvant être modulé par l'autorité organisatrice de transports. Les entreprises de transport auraient été tenues de requérir les personnels nécessaires pour assurer ce service minimal, sous peine d'amende administrative. Sur ma proposition, la commission a adopté un amendement visant à assurer la constitutionnalité et le caractère

Les réalités ne sont, en effet, pas les mêmes d'un territoire à l'autre, selon qu'il existe ou non des alternatives aux transports publics. Lorsque l'offre de transports publics est diversifiée, par exemple en zone urbaine, il convient d'adopter une approche globale. La commission a en outre relevé que l'application de la règle de l'arrondi à l'entier supérieur conduirait en pratique, lorsqu'il n'existe que quelques dessertes par jour, à un niveau de service nettement supérieur à un tiers Dès lors, restreindre le droit de grève sans l'adapter aux besoins réels de la population pourrait constituer une atteinte excessive à un droit de valeur constitutionnelle. Une telle proposition encourrait très probablement la censure du Conseil constitutionnel. L'article 3, tel que récrit par la commission, laisse donc aux autorités organisatrices de transports, c'est-à-dire, le plus souvent, aux régions ou aux intercommunalités, le soin de définir au cas par cas le niveau minimal de service nécessaire. Cette définition prendrait la forme d'une délibération, susceptible d'être déférée devant le juge administratif. Par hypothèse, une situation dans laquelle ce niveau minimal ne serait pas assuré constituerait une atteinte à la satisfaction des besoins de la population et autoriserait une limitation du droit de grève. Toutefois, considérant que la population a une capacité d'adaptation, et dans le souci d'apporter au droit de grève une limitation proportionnée, la commission a prévu un délai de carence de trois jours, à l'issue duquel l'autorité organisatrice de transports pourrait enjoindre aux entreprises concernées de requérir les personnels nécessaires. Un salarié qui refuserait de se conformer à l'ordre de son employeur formulé dans ce cadre ferait alors un usage illicite de son droit de grève et serait donc passible de sanctions disciplinaires. L'article 6 prévoit des dispositions relatives au remboursement des usagers qui n'ont pas pu voyager. Les transporteurs proposent bien souvent un échange ou un avoir, alors que les usagers sont en droit d'attendre un remboursement, de préférence sans avoir à en faire la demande. La commission a adopté cet article en lui apportant des modifications rédactionnelles. Le texte étend par ailleurs aux liaisons maritimes de desserte des îles françaises les dispositions de la loi de 2007 et celles introduites par la proposition de loi. La commission a complété ces dispositions pour que s'appliquent à ces liaisons l'ensemble des dispositions du code des transports relatives à la prévention des conflits collectifs et à l'encadrement du droit de grève. grève. L'article 8 concerne le secteur aérien. Sur ma proposition, la commission a adopté un amendement tendant à limiter l'application du dispositif aux seules lignes sous obligation de service public, soit une douzaine de lignes en France continentale ainsi que certaines liaisons entre la Corse et le continent et entre la métropole et les outre-mer. Elle a ainsi établi une symétrie avec les dispositions de l'article 3, qui ne visent que les services publics de transport terrestre, et mis le dispositif en conformité avec le droit européen qui régit le secteur. La commission a par ailleurs renforcé la possibilité pour les compagnies aériennes de réorganiser le service en utilisant les déclarations individuelles d'intention de faire grève, la Cour de cassation ayant jugé que le droit actuel ne le permettait pas. La commission a également complété cette proposition de loi par des dispositions de nature à lutter contre certains abus constatés en matière d'exercice du droit de grève qui pénalisent indûment les usagers. Si la procédure d'alarme sociale introduite par la loi de 2007 a permis d'améliorer le dialogue social et de réduire la conflictualité dans les transports publics, on observe pourtant des stratégies visant à contourner cette obligation de négociation et même l'obligation de préavis. Il n'est pas rare que des organisations syndicales déposent des préavis très longs ou illimités sur des sujets très larges, comme les salaires ou les conditions de travail. Ces préavis demeurent en vigueur même si le conflit a cessé, si bien qu'à tout moment des salariés peuvent se mettre en grève en n'ayant à respecter que le délai de prévenance de quarante-huit heures. Il s'agit là d'un contournement manifeste de la loi de 2007. Aux termes de l'article 9 introduit par la commission, un préavis de grève pourra être déclaré caduc par l'entreprise dès lors qu'il n'aura été suivi par aucun salarié pendant une période de cinq jours. Cette mesure n'entrave pas la liberté des organisations syndicales, qui pourront toujours appeler à la grève dès lors qu'elles l'estimeront nécessaire, en respectant les règles. La commission a également ajouté un article 10 visant à lutter contre les grèves de très courte durée, dites « de 59 minutes », qui désorganisent fortement les réseaux de transport. Un conducteur de bus ou de tramway qui a décidé de se mettre en grève pendant une heure au milieu de son service oblige son employeur à le remplacer pour l'intégralité de ce service, sans qu'il soit nécessairement possible de le réaffecter lorsque sa grève prend fin.

Voilà, mes chers collègues, le sens des modifications que nous avons apportées à la proposition de loi. Nous en avons conservé tous les objectifs et n'en avons modifié les contours, avec l'accord de ses auteurs, que pour sécuriser ses dispositions. La commission des affaires sociales vous demande de l'adopter. La parole est

entre le 5 décembre et le 17 janvier derniers, les Françaises et les Français ont subi six semaines d'une grève de grande ampleur dans les transports, notamment en Île-de-France. Cette grève a eu des conséquences importantes pour bon nombre de nos compatriotes, qu'ils soient salariés, étudiants ou retraités. L'allongement des temps de transport a conduit beaucoup de Français à se lever très tôt le matin et à rentrer chez eux tard le soir pour respecter au mieux leurs horaires de travail. De nombreuses entreprises ont vu leur activité perturbée et des interventions médicales ou des examens universitaires ont dû être aménagés ou reportés. La continuité du service de transport de voyageurs est essentielle à la vie quotidienne des Français et à l'activité économique du pays. Je comprends Je comprends donc que le Sénat ait souhaité, par la voix du président du groupe majoritaire, Bruno Retailleau, faire évoluer de manière substantielle le cadre juridique dans lequel s'exerce le droit de grève dans les transports publics, en instaurant une véritable garantie de service minimum. Je peux même dire que je partage l'objectif ultime des auteurs du texte, qui est d'assurer la continuité du service public et de permettre l'exercice dans les faits du « droit à la mobilité ce droit que nous avons choisi d'inscrire, il y a peu, en ouverture du code des transports et dont nous souhaitons qu'il soit effectif pour tous, au quotidien, dans tous les territoires. Dans le même temps, le Gouvernement est profondément attaché au respect du droit de grève, constitutionnellement garanti par le Préambule de la Constitution de 1946. Vous l'avez dit, monsieur Retailleau : il revient au législateur d'accomplir la tâche difficile de conciliation de ce droit avec le principe de continuité du service public.

Pour autant, l'épisode de ces derniers mois met en lumière les limites de notre cadre actuel, et il est légitime que la représentation nationale se saisisse du sujet. Pour aller plus loin, il me semble toutefois indispensable de disposer d'une analyse juridique approfondie et de se laisser le temps de la concertation avec les parties concernées. indispensable, car l'instauration d'un service minimum dans les transports implique de concilier plusieurs objectifs de valeur constitutionnelle. Or la rédaction actuelle de la proposition de loi me semble fragile sur le plan juridique et présente un risque réel de censure par le juge constitutionnel.

Dans ces conditions, l'encadrement du recours au service minimum par les autorités organisatrices apparaît insuffisant pour garantir la constitutionnalité du dispositif. du dispositif. Les questions juridiques sont donc nombreuses et méritent d'être approfondies au-delà du travail de grande qualité accompli par Mme la rapporteure Pascale Gruny. Il convient également de progresser dans l'articulation avec les dispositions existantes, notamment celles de la loi de 2007. de la loi de 2007. Il me semble en outre nécessaire de prendre le temps de la concertation sociale. La grève qui bloquait les transports collectifs s'est arrêtée courant janvier et le contexte commande désormais l'apaisement des relations avec le corps social des entreprises concernées. Partageant toutefois l'esprit qui vous anime, mesdames, messieurs les sénateurs, et puisque le Gouvernement doit sécuriser le dispositif avant de pouvoir envisager de l'inscrire dans notre droit, je propose de lancer dans les prochaines semaines une mission sur ce thème. Pilotée par un juriste éminent qui pourrait être issu du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, celle-ci devra faire des propositions sous deux mois, afin que nous en puissions en disposer pour la suite du débat parlementaire. Cette mission portera sur les conditions de l'installation d'un service minimum garanti dans les transports, mais également sur les deux autres points que vous soulevez au travers de votre proposition les préavis illimités, d'une part, et, d'autre part, les grèves de très courte durée, dites « grèves de 59 minutes », qui, nous le savons, perturbent gravement l'organisation du service. Ses conclusions nous permettront d'appréhender le sujet de manière sécurisée et de travailler à un dispositif qui devra être à la fois constitutionnel et opérationnel.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi, sous couvert d'assurer l'effectivité du droit au transport, porte une atteinte grave au droit de grève, constitutionnellement garanti par les jurisprudences du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État et de la Cour de cassation. À vrai dire, nous ne sommes pas surpris de cette initiative, dont l'objet « signaler » aux usagers des transports en commun qu'en soutenant massivement le mouvement de grève de ces dernières semaines, ils n'ont en fait rien compris : en réalité, la grève, ça les dérange, et la droite sénatoriale va régler ça

à 1 500 euros ! Par ailleurs, comment ne pas voir de vraies convergences d'intérêts entre les grévistes et les usagers ? En effet, toutes les dernières grèves dans le secteur des transports se donnaient pour objectif la défense du service public, et donc l'intérêt des usagers, face aux velléités de démantèlement et de libéralisation. Votre vote du pacte ferroviaire et de la loi d'orientation des mobilités (LOM) entraîne en effet directement la dégradation du service et la galère quotidienne pour l'ensemble des usagers, celle-là même que vous dénoncez aujourd'hui.

le contexte particulier dans lequel ce texte est débattu. Est-ce là la réponse de la majorité sénatoriale au rejet massif de la réforme des retraites ? Dans une situation de tension sociale majeure, où un pouvoir « droit dans ses bottes » remet en cause les fondements du pacte républicain issu du programme du Conseil national de la résistance, votre groupe s'attaque aux grévistes pour les contraindre à rentrer dans le rang en courbant l'échine. Vous vous en prenez aujourd'hui aux transports de personnes, mais j'ai le sentiment que votre ambition est plus large. Ce que vous voulez, c'est bel et bien retirer aux salariés le droit ultime dont ils disposent pour défendre leurs intérêts, les laissant vulnérables et impuissants dans la guerre sociale menée par ce gouvernement ne faut pas exagérer ! Ce faisant, vous êtes les alliés de ce pouvoir rétrograde que vous ne manquez pas de vilipender quand cela vous arrange

! Eh oui ! Les tentatives de la commission pour « border » un texte inacceptable ne masquent pas un véritable aveu de culpabilité s'agissant du caractère inconstitutionnel de ce texte. Nous regrettons d'ailleurs de ne pas disposer d'un avis du Conseil d'État. Porter atteinte au droit de grève pour l'ensemble des transports de personnes, maritimes, terrestres et aériens, ne peut se faire à la hussarde, sans éléments juridiques tangibles. exposé des motifs est à ce titre assez fascinant. Il évoque pêle-mêle la liberté d'aller et venir et la liberté du travail comme principes qui justifieraient des restrictions au droit de grève.

contrairement au droit au travail, défini comme un droit social garanti par le Préambule de la Constitution de 1946. L'exposé des motifs mentionne également la « liberté d'accès au service public », alors que les principes reconnus par la jurisprudence sont ceux d'« égal accès aux services publics » et de « continuité du service public ». Pourquoi autant d'inepties ? Si nous nous référons bien aux mêmes principes constitutionnels, la seule conciliation dont nous pouvons convenir recherchée entre le droit de grève et le principe de continuité des services publics. Dans ce cadre, il existe une jurisprudence à laquelle il convient de se référer.

que « ces limitations [ne] peuvent aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents » que pour ceux « dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ». Ce n'est quand même pas la même chose

D'ailleurs, le rapport Mandelkern du Conseil d'État, base du projet de loi de 2007, reconnaissait lui-même l'existence d'une très grande incertitude sur ce point. Les auteurs de ce rapport notaient également que l'interdiction du droit de grève sur le fondement des « besoins essentiels du pays » doit être limitée au strict nécessaire. Tel n'était pas le cas dans le texte initial de cette proposition de loi, qui prévoyait le maintien d'un tiers du trafic. On était bien loin de cette « stricte nécessité », et même du principe de proportionnalité, également reconnu par le Conseil constitutionnel lorsqu'il est porté atteinte à un droit de valeur constitutionnelle. l'instauration d'une carence de trois jours avant le recours à la réquisition n'est pas de nature à garantir cette stricte proportionnalité. Par ailleurs, le choix fait par la commission, pour éviter cet écueil, de renvoyer la définition des services essentiels, et donc du niveau de réquisition, aux autorités organisatrices reste problématique. Rien ne garantit que certaines autorités ne feront pas le choix d'un service minimum allant au-delà du tiers des dessertes initialement prévu. En outre, nous estimons qu'il s'agit d'un jeu dangereux. Que les autorités organisatrices exercent leur compétence en matière de transports, c'est une chose ; en faire des des acteurs du rapport de force qui s'établit dans le cadre d'un mouvement social, c'est autre chose. Il n'est d'ailleurs pas certain que les élus souhaitent endosser cette responsabilité sociale de facilitateur ou de censeur de grève.

Le droit de grève ne peut souffrir cette « balkanisation ». Il faut rappeler que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 juillet 1980,

droit. Cette même décision indique également que la loi ne saurait comporter aucune délégation au profit du Gouvernement, de l'administration ou de l'exploitant du service en matière de réglementation du droit de grève. Ainsi, laisser aux autorités organisatrices le soin de définir les services essentiels et à l'entreprise l'exercice de la réquisition est manifestement inconstitutionnel. Par ailleurs, ce dispositif, qui vise à organiser la mise en place de dessertes garanties, soulève le problème de la traduction de la multiplicité des rapports des pouvoirs locaux par la multiplicité des conditionnements du droit de grève et des inégalités dans son exercice, liée notamment à la difficile ouverture à la concurrence des transports régionaux. Vous l'aurez compris,

est un signe de faiblesse, et non de force. Cessez de jouer les pompiers pyromanes ! Pour réduire la conflictualité sociale, demandez avec nous le retrait du projet de loi de réforme des retraites. Vous verrez, tout rentrera dans l'ordre ! Demandez avec nous l'instauration d'un dialogue social respectueux des syndicats ! Exigez enfin le maintien et le développement du service public afin de garantir aux usagers fiabilité, confort et sécurité ! En conclusion, je vous serais reconnaissante de ne pas convoquer Maurice Thorez, sauf à citer l'intégralité de ses propos : « Il faut savoir terminer une grève dès que la satisfaction a été obtenue. Il faut même savoir consentir au compromis si toutes les revendications n'ont pas encore été acceptées mais que l'on a obtenu la victoire

la formule républicaine a su admirablement ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait ; la gradation [ ...] est irréprochable. Liberté, Égalité, Fraternité. Rien à ajouter, rien à retrancher. Ce sont là les trois marches du perron suprême. La liberté, c'est le droit, l'égalité, c'est le fait, la fraternité, c'est le devoir. Tout l'homme est là. » Voilà ce que disait le plus illustre des sénateurs, Victor Hugo, sur la devise de notre pays. C'est à la lumière de ces mots que je souhaite examiner la proposition de loi, présentée par Bruno Retailleau et de très nombreux collègues, visant « à assurer l'effectivité du droit au transport, à améliorer les droits des usagers et à répondre aux besoins essentiels du pays en cas de grève La liberté, c'est le droit. Le droit de grève en France est un droit à valeur constitutionnelle, et personne ne le conteste. Le droit à la continuité des services publics est également un droit à valeur constitutionnelle.

que nous examinons aujourd'hui est donc de débloquer une situation devenue insupportable, tout en respectant scrupuleusement ces droits fondamentaux et leur valeur constitutionnelle. C'est tout simplement un véritable rééquilibrage des droits qu'il est proposé de mettre en oeuvre ici. On est donc aux antipodes de l'exception d'irrecevabilité invoquée par nos collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. En effet, la liberté d'aller et venir est une composante fondamentale de la liberté individuelle. Chacun peut circuler sur l'ensemble du territoire national dès lors qu'il y est régulièrement Or, pendant plus d'un mois, cette mission de service public n'a plus été assurée normalement dans notre pays. Dans ces conditions, garantir un trafic quotidien constitue non pas un recul des droits fondamentaux, mais plutôt le strict minimum pour que la liberté de chacun soit respectée. L'égalité, c'est le fait. En 2020, mes chers collègues, on est en droit d'attendre que l'exercice d'un droit de grève mature puisse, certes, perturber un service public, mais en aucun cas le bloquer totalement Il n'est en effet plus possible que le droit de grève conduise une minorité organisée à prendre tout un pays et toute une économie en otage. C'est vrai ! Ce n'est C'est pour éviter cette paralysie qu'est proposée la création d'un service minimum de transport garanti applicable aux transports publics ferroviaire, aérien et maritime. C'est bien de cela qu'il s'agit dans cette proposition de loi, et non pas d'une quelconque remise en cause liberticide d'un droit fondamental. Le futur service minimum garanti contribuera ainsi à assurer la liberté d'aller et venir, la liberté d'accès aux services publics, la liberté du travail- n'en déplaise à certains ! -, la liberté du commerce et de l'industrie, tout en préservant la liberté de faire grève. La loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs a constitué indéniablement un progrès, mais, reconnaissons-le, elle n'a pas permis d'atteindre l'objectif d'assurer, en toutes circonstances, la continuité du service public. Pourtant, comme le rappelle fort justement notre collègue Pascale Gruny dans son rapport, la jurisprudence du Conseil constitutionnel prévoit la possibilité d'interdire purement et simplement le droit de grève aux agents « dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services publics dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays

je crois que nous pouvons raisonnablement estimer que les transports publics correspondent aussi à un « besoin essentiel du pays ». La fraternité, c'est le devoir. La loi du 21 août 2007 prévoit des règles pour favoriser le dialogue social et permettre une meilleure organisation des services de transports publics en cas de grève. Elle instaure l'obligation pour les salariés d'indiquer quarante-huit heures à l'avance leur intention de faire grève. La mise en oeuvre d'un service minimum aux heures de pointe est laissée aux accords entre syndicats et autorités organisatrices. Cette première étape de négociation est indispensable, et elle doit demeurer. En revanche, lorsqu'elle s'avère inopérante, un dispositif complémentaire doit permettre d'assurer la continuité du service public de transport. Tel est l'objet de la présente proposition de loi, qui s'attache à rendre obligatoire le fonctionnement partiel des transports publics les jours de grève. Il s'agit, enfin, de partir des besoins de la population et d'en assurer la couverture, et non pas de partir du nombre de grévistes pour prévoir le service qui peut être assuré. Cela paraît tout de même évident Alors peut-être en finirons-nous enfin avec ces agressions dévastatrices entre grévistes et non-grévistes, entre ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler et ceux qui s'y opposent parce qu'ils revendiquent et qui voudraient créer le chaos alors que notre nation a besoin d'unité N'oublions pas que les premières victimes des mouvements de grève dans les transports, ce sont nos concitoyens les plus fragiles économiquement, comme l'a dit Bruno Retailleau, ceux qui n'ont pas les moyens de recourir à des solutions de repli. Il s'agit des salariés qui résident loin de leur lieu de travail et ne disposent pas d'un véhicule personnel, de ceux qui ne bénéficient pas d'une autonomie professionnelle leur permettant d'adapter leurs horaires de travail ou de télétravailler eux qui ont été les plus touchés ! Par ailleurs, mes chers collègues, il y a une nouvelle donne que nous devons absolument prendre en compte : je veux parler de l'enjeu écologique La substitution du transport collectif au transport individuel est l'une des réponses essentielles aux enjeux environnementaux. Les cars Macron ! En ce domaine, la France a encore beaucoup de progrès à faire puisque, dans un jugement du 24 octobre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que notre pays avait dépassé depuis 2010 « de manière systématique et persistante » le seuil limite de dioxyde d'azote, un gaz produit notamment par les moteurs diesel. Ce jugement pourrait conduire, dans un deuxième temps, à des sanctions si la France ne faisait rien pour remédier à cette situation. Nous sommes tous d'accord pour dire que le développement du transport collectif est une des solutions pour remédier à ces mauvais résultats. lors, il doit être encouragé et accéléré. Il le sera d'autant plus que les transports publics apparaîtront enfin fiables et assurant en toutes circonstances le transport des passagers. On ne peut pas à la fois promouvoir les vertus du transport public et ne pas lui imposer des obligations de régularité de service. Cela paraît, là encore, assez évident La place des transports publics croît dans les habitudes de déplacement des Français. Dans son dernier rapport, remis en 2019, le Commissariat général au développement durable a indiqué que la France était passée, pour ce qui concerne le transport collectif, de 152,4 à 200 milliards de voyageurs-kilomètres entre 2001 et 2016. Cette progression souligne l'importance des transports collectifs dans la vie quotidienne de nombreux Français. Le respect de la continuité du service public de transport est une des conditions indispensables de sa croissance rapide. Comment ne pas évoquer également les problèmes de santé publique causés par les difficultés de circulation ? Le porte-parole Le porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris a fait état d'une hausse de 40 % des accidents constatés dans la capitale, notamment pour les deux-roues. Les embouteillages ont provoqué des retards d'intervention des véhicules de pompiers et de secours. C'est la faute des grévistes ? Les hôpitaux ont également signalé l'augmentation des pathologies liées à la pollution et une baisse

Ces mesures vont de l'autorégulation, avec l'accord des partenaires sociaux, dans les pays du Nord, à la réquisition des personnels en Grande-Bretagne, ou même à la garantie d'un service normal dans les transports en Italie. Notre pays se distingue donc une fois de plus par son inaction. Qu'attendons-nous, monsieur le secrétaire Après la liberté, l'égalité, la fraternité, l'écologie et la santé, permettez-moi d'évoquer un nouveau paramètre de la grille de lecture : la justice.

En effet, si la SNCF et la RATP sont incapables, nonobstant leur monopole, d'assurer un service digne de ce nom, elles s'avèrent en revanche beaucoup plus expertes quand il s'agit de débiter avidement les comptes des usagers dont le voyage est annulé tout en osant leur proposer un avoir

C'est bien la moindre des choses ! Monsieur le secrétaire d'État, il est maintenant de votre responsabilité de prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la continuité effective du service de transport de voyageurs et de marchandises. Forts de notre expérience d'élus confrontés aux troubles de l'ordre public sur nos territoires, nous vous proposons ici un dispositif équilibré, proportionné, efficace et respectueux des droits de chacun

Au demeurant, nous ne sommes pas d'accord avec les arguments juridiques avancés par ses auteurs. Le Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Par ces mots, le constituant a tout à la fois conféré une valeur constitutionnelle au droit de grève, ce que nul ici ne conteste, et affirmé que le législateur était compétent pour définir les limites qu'il convient d'apporter à ce droit,

conformer aux différentes stratégies gouvernementales, qu'il s'agisse de la stratégie nationale bas carbone ou de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Sur le plan des faits, je voudrais souligner que,

Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? ... Je mets aux voix la motion n° 5, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet de la proposition de loi.

chers collègues, la grève, comme le disent ces vers puissants de Jacques Prévert, constitue l'ultime moyen dont disposent les travailleurs pour faire face à une attaque contre leurs droits, n'en déplaise à certains. Ils n'ont sûrement pas à rougir de son exercice, car ils sont bien dans leur droit, celui de défendre des conquis sociaux, issus de grandes luttes. Aujourd'hui, ce sont nos retraites qui sont remises en cause par le patronat, avec l'appui du gouvernement en place. Au lieu de fustiger, comme vous le faites au travers de cette proposition de loi, les agents des transports grévistes et de les traiter comme des preneurs d'otages, nous devrions tous et toutes et toutes les remercier de défendre notre système solidaire de retraites par répartition contre un gouvernement souhaitant voir les salariés travailler à vie et les dépouiller au profit de

contre le désengagement de l'État et la privatisation qui entraînent la dégradation de ceux-ci et les difficultés quotidiennes rencontrées par nos concitoyens pour se déplacer.

qui vise, une fois encore, à restreindre le droit de grève des agents des transports publics. Devons-nous encore vous rappeler que l'effectivité du droit au transport, si cher à vos coeurs, vous l'avez vous-mêmes enterrée en votant toutes les lois de démantèlement du service public ? Je ne reviendrai pas sur l'inconstitutionnalité d'un tel dispositif, qui va jusqu'à prévoir la réquisition des grévistes, comme l'a si bien démontré ma collègue Éliane Assassi, mais je souhaite insister sur un point fondamental d'opposition entre nous : notre conception du service public des transports n'est sûrement pas la même que la vôtre. Nous nous battons aux côtés des agents des transports publics et de leurs organisations syndicales pour un véritable service public de qualité et de haut niveau pour tous les usagers. Je vous renvoie à ce titre au débat sur la réforme ferroviaire qui nous a opposés sur ces travées. Lutter pour un véritable service public nécessite d'abord de revenir sur les politiques de libéralisation et de privatisation de nos entreprises publiques de transport. il s'agit de redonner des moyens financiers et humains au secteur des transports, dont l'État n'a eu de cesse, depuis des décennies, de se désengager, avec votre soutien. Ces logiques ont conduit à des drames. Ce fut le cas avec l'accident ferroviaire de Brétigny, causant 7 morts et plus de 400 blessés, alors que les représentants du personnel avaient alerté à maintes reprises leur direction sur le risque d'une catastrophe.

la grève ou de tout autre conflit. Or dans le cadre d'une société capitaliste, le conflit est intrinsèquement lié à l'antagonisme des intérêts entre capital et travail. La grève est un moyen de rééquilibrer le rapport de force en faveur des salariés, mais vous souhaitez la faire disparaître, ... Non ! ... y compris en usant de la force, comme avec la réquisition. Or, en faisant cela, vous donnez encore davantage de pouvoir à l'employeur qui, en plus de détenir le pouvoir de dégrader les conditions de travail de ses salariés, pourra anéantir toute forme d'expression conflictuelle tendant à rééquilibrer la relation de travail, par nature inégalitaire. Il s'agit là d'une attitude irresponsable et d'une entreprise dangereuse, surtout lorsqu'elle se pare des meilleures intentions, comme c'est le cas avec votre texte. Nous observons en effet depuis de nombreuses années, et encore dans le cadre du mouvement social actuel, un accroissement de la répression syndicale, avec une volonté, de la part des directions des entreprises de transport, mais aussi du Gouvernement, de museler les agents refusant d'accompagner les politiques de privatisation et de dégradation tant du service public que de leurs conditions de travail. Vous trompez également les usagers en leur faisant croire que les difficultés rencontrées au quotidien sont dues aux mouvements de grève. On rêve ! De plus, le droit de grève n'appartient pas seulement aux agents de transports mais à tous les salariés, dont les usagers des transports. Autrement dit, vous vous attaquez de fait aux droits des usagers et de tous les salariés dans leur ensemble. Pour ces raisons,

grève par procuration, grève perlée, grève tournante, grève surprise, grève de solidarité ... La grève sous toutes ses formes ! Il y a ceux qui la font et ceux qui peuvent être amenés à la subir. Il existe cependant d'autres droits, tout à fait objectifs, et nous devons respecter le fait qu'un droit ne doit pas prendre le pas sur un autre. Nous avons vu ces derniers mois le droit de grève faire échec à la liberté d'aller et venir, à la liberté du commerce et de l'industrie, à la continuité du service public. Les PME ont particulièrement souffert de l'absence de leurs salariés. Eux-mêmes ne peuvent souvent pas faire grève, sauf à risquer de perdre leur emploi. Comment admettre que des salariés se retrouvent aujourd'hui au chômage à la suite du dépôt du bilan de leur entreprise, incapable d'exercer ses activités ? Les transports publics sont en effet essentiels à l'exercice de bon nombre de nos libertés. Beaucoup de nos concitoyens ont ainsi été dans l'impossibilité de se rendre sur leur lieu de travail. Beaucoup de commerces ont connu une faible fréquentation au moment qui aurait dû être le plus favorable pour eux en termes de chiffre d'affaires. La grève est plurielle. Il y a celle qui a pour objet d'appuyer des revendications professionnelles dont la satisfaction dépend de l'employeur. C'est alors un outil de négociation dans les conflits du travail. Mais il est aussi des grèves qui appuient des revendications professionnelles dont la satisfaction ne dépend nullement de l'employeur.

qui n'ont pas le pouvoir de retirer un projet de réforme. C'est à la démocratie de trancher ces sujets. Nous assistons ainsi parfois à des abus abus du droit de retrait, derrière lequel la grève peine à se dissimuler ; abus de l'exercice du droit de grève lui-même, chaque fois qu'il est détourné de sa finalité ou que les conditions de sa légalité ne sont pas respectées. C'est le cas aussi lorsque la grève se transforme en un instrument de pression sur des salariés non grévistes ces pressions sont illégales et inacceptables. La grève est un droit dont l'exercice doit respecter les formes prescrites et ne pas mettre en péril le nécessaire équilibre entre les différents droits et libertés de valeur constitutionnelle.

Le droit de grève peut être et doit être encadré afin de contenir d'éventuelles conséquences disproportionnées. Cela a déjà été fait par la loi de 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.

Ce préavis est essentiel. C'est pourquoi nous vous proposons d'étendre cette obligation aux contrôleurs aériens. Le groupe Les Indépendants avait déposé une proposition de loi en ce sens ; je vous suggère aujourd'hui de voter par amendement le dispositif adopté en commission. Car rares sont ceux qui savent que les contrôleurs aériens ne sont pas soumis à un préavis La loi de 2007 ne permet cependant pas d'empêcher les situations de paralysie, quand les revendications professionnelles ne dépendent pas de l'employeur. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à établir un service minimum effectif, afin de satisfaire aux besoins essentiels de la population.

Celle-ci ne trouvera à s'appliquer que lorsqu'elle est strictement nécessaire à la satisfaction des besoins essentiels de la population. Nous devons cependant veiller à ce que cette nouvelle prérogative ne soit pas porteuse de risques juridiques pour les collectivités de nos territoires, mais aussi à ce que les collectivités à ce que les collectivités n'aient pas à suppléer d'éventuelles carences de l'État, comme ce fut le cas avec la loi Darcos, qui oblige les communes à assurer un service minimum d'accueil des enfants en cas de grève dans l'éducation nationale.

Nous sommes également convaincus que cela pourrait susciter des échanges respectueux et constructifs entre les usagers et les grévistes, sortant de la logique d'affrontement. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants soutient et approuve cette proposition de loi, tout en restant attentif au respect des équilibres entre les différents droits et libertés. La parole est à Mme Jocelyne Guidez. Madame

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi tendant à assurer l'effectivité du droit au transport, à améliorer les droits des usagers et à répondre aux besoins essentiels du pays en cas de grève. Je tiens à saluer l'initiative des auteurs de cette proposition de loi, ainsi que notre rapporteur tant pour son travail très approfondi que pour les précisions juridiques qu'elle a apportées en commission. Le préambule de la Constitution de 1946 énonce : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale [ ...] ». La grève est une des actions possibles. Mais ce préambule prévoit aussi que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent et c'est là tout l'objet de la présente proposition de loi. Il est incontestable et incontesté que, historiquement, certaines grèves ont permis aux travailleurs, puis à l'ensemble de la population, d'obtenir bon nombre de droits sociaux fondamentaux. Ce faisant, la grève a indéniablement participé à la construction de l'État-providence. Aujourd'hui, de nombreuses grèves n'opposent plus les employés aux employeurs, mais constituent un levier d'action pour manifester contre la politique du Gouvernement.

Par ailleurs, il affecte directement les usagers des transports publics, mais aussi tout un pan du monde économique, dont les activités dépendent du ferroviaire, du maritime ou des transports aériens. Plus singulièrement, les transports publics subissent inévitablement les effets collatéraux de certains mouvements de grève. Mais pas seulement eux ! Certains acteurs économiques ont été particulièrement touchés par ces grèves, qu'il s'agisse d'entreprises ou de commerces. Surtout, ces derniers subissent régulièrement les effets de mouvements sociaux de grande ampleur, qui fragilisent leur santé financière, et, dans le pire des cas, ils sont contraints de licencier des salariés, voire de cesser leur activité. C'est pourquoi cette proposition de loi prend acte d'un constat : malgré la valeur constitutionnelle de ces deux normes, l'équilibre entre le droit de grève et le principe de continuité a basculé en faveur du premier. Un nécessaire rééquilibrage est juridiquement réalisable, conformément à la position du Conseil constitutionnel sur le sujet. C'est ainsi que cette proposition de loi s'inscrit pleinement dans la continuité de la loi du 21 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Précisément, cette proposition de loi vise à ce que l'autorité organisatrice de transport (AOT) définisse, par une délibération publique transmise au préfet, un niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population. Ce n'est que dans le cas où un minimum de service ne serait pas assuré pendant une durée de trois jours consécutifs que l'AOT pourrait demander à l'entreprise de transport de recourir à la réquisition des personnels indispensables pour assurer le niveau minimum de service. L'entreprise aura alors l'obligation de se conformer à cette injonction dans un délai de Des dispositions similaires concernent les transports maritimes réguliers publics de personnes outre-mer et les services aériens réguliers. Par exemple, en janvier 2020- ce n'est pas si ancien en raison de fortes grèves chez les dockers, la Martinique et d'autres îles n'ont pas pu être approvisionnées en produits alimentaires et de première nécessité. Tout à fait ! N'est-ce pas prendre toute une population en otage ? Cette proposition vient donc compléter la loi de 2007. Elle est une réponse apportée aux victimes de l'échec des négociations préalables à la grève. Il nous paraît aujourd'hui juridiquement possible et socialement souhaitable de préciser les contours du droit de grève., il s'agit de permettre aux salariés de défendre leurs droits, tout en garantissant aux personnes lésées par la grève que les leurs ne seront pas, outre mesure, affectés. C'est pourquoi la majorité des membres du groupe Union Centriste soutiendra cette proposition de loi. Bravo ! La parole

d'État, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui a été déposée le 2 décembre, au début d'un mouvement d'ampleur inédite dans les transports contre le projet de réforme des retraites. Cette proposition de loi est incontestablement une proposition d'affichage politique, un petit coup de pied de l'âne aux syndicats qui préparaient une journée d'action pour le 5 décembre dernier, et une manière à mon sens peu délicate d'anticiper, voire d'attiser, des conflits des conflits d'intérêts divergents entre les grévistes et les usagers. Par ailleurs, vous avez sans doute observé, comme moi, que si les usagers, dont les témoignages ont été recueillis quasi quotidiennement par les médias tout au long du mouvement sur les quais des gares et du métro, ont accueilli avec un soulagement non dissimulé le retour des trains et des métros à la circulation, peu d'entre eux se sont laissés aller jusqu'à remettre le droit de grève en question. C'est pourtant ce que les auteurs de cette proposition de loi n'hésitent pas à faire. celle-ci aurait tout aussi bien pu s'intituler « proposition de loi pour limiter le droit de grève dans les transports par la réquisition des personnels » : cela aurait été assez conforme à son objet, car le coeur de ce texte est un transfert et un élargissement du droit de réquisition. La proposition de loi opère plusieurs ruptures importantes avec le droit positif. Rappelons que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, que le législateur, ainsi que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, a d'encadrer pour le concilier avec un autre principe constitutionnel : la sauvegarde de l'intérêt général. Ce souci de conciliation entre deux principes pouvant se contrarier a déjà conduit à un encadrement du droit de grève, qui peut aller parfois jusqu'à l'interdiction de ce droit, lorsque la grève porte atteinte aux besoins essentiels du pays. Ces restrictions légales sont précises et visent à protéger l'ordre public. Le code de la santé, par exemple, prévoit que, pour faire face à un afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, le représentant de l'État peut requérir toute personne nécessaire. Aujourd'hui, au moment même où nous parlons, le préfet d'Île-de-France a requis,

Personne ne conteste que la grève occasionne de nombreux désagréments aux usagers. Mais elle ne crée ni un trouble à l'ordre un trouble public ni une situation de crise. Nous ne sommes pas allés jusque-là ! Votre proposition d'étendre à des entreprises privées, privées, nombreuses dans les transports, un droit de réquisition qui est aujourd'hui une prérogative de l'État par l'intermédiaire des préfets vise, en fait, à privatiser le droit de réquisition. Cette privatisation est plus qu'un glissement, c'est une dérive, et une dérive grave, car le droit de réquisition doit demeurer strictement régalien. L'article 3 fait peser sur les entreprises de transport une obligation de service minimum, assortie de pénalités financières en cas d'impossibilité d'atteindre cette obligation de résultat, sans qu'il soit dit comment ces entreprises pourront faire respecter cette obligation. Vous prévoyez une sanction disciplinaire. Pourtant, vous savez tous, sans doute, que la Cour de cassation a déclaré en 2009 qu'un gréviste ne pouvait pas être sanctionné en raison de son refus d'obtempérer à une réquisition. les conséquences sur le droit du licenciement, sur les travailleurs à statut, les salariés de droit privé, le code du travail ... ? On ne sait pas ! Tout cela n'est pas très sérieux et prouve, à mon sens, que cette proposition de loi est d'abord un texte de propagande politique, qui consiste à faire de l'exception le droit courant, le droit commun. Ce texte prévoit que la réquisition des salariés, grévistes ou non, deviendrait la procédure systématique applicable à toutes les grèves dans les transports. Il instituerait ainsi un droit de grève restreint pour les agents et les salariés des transports. Or ce qui est nécessaire pour le maintien de l'ordre public dans le secteur de la défense ou dans les hôpitaux ne peut être systématiquement et transposable aux activités des transports. La loi de 2007 a favorisé le dialogue social, tous les acteurs en conviennent aujourd'hui. Votre proposition de loi ne favoriserait que le conflit, dans l'entreprise comme entre les usagers et les grévistes. Elle constituerait un recul grave en matière de libertés publiques et un précédent dans la restriction des droits des salariés à défendre et leurs conditions de travail et la qualité du service public. En effet, je considère que, lorsque les agents et les salariés d'un service défendent leurs conditions de travail, ils défendent aussi la qualité du service aux usagers. Quant à l'argument, développé par le président Retailleau,

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, avec la proposition de loi de nos collègues du groupe Les Républicains, nous nous penchons sur une question éminemment sensible, celle du droit de grève et des restrictions que nous pouvons ou pas lui apporter. Une fois n'est pas coutume, notre groupe, riche de sa diversité, ne se positionnera pas de façon unanime. Chacun votera selon ses convictions, et c'est avec les miennes que je m'exprime devant vous. Avant d'aborder le contenu même du texte, on peut légitimement soulever un préalable la période est-elle la plus opportune pour en débattre, alors que les perturbations issues des grèves contre la réforme des retraites ont hystérisé la situation ? C'est un sujet grave, mettant en jeu l'une nos libertés publiques fondamentales et fondatrices. nous devons donc d'aborder ce type de réflexion dans le calme et dans un climat apaisé, détachés, les uns et les autres, des émotions que nous avons pu vivre ces dernières semaines ... Des émotions nécessairement affectées par nos situations individuelles, selon, par exemple, que l'on est francilien ou provincial, usager ou non des transports en commun. Sur le sujet précis de l'encadrement du droit de grève, nos réflexions doivent être guidées, il me semble, par deux principes que j'estime fondamentaux : la nécessité et la proportionnalité. En d'autres termes, notre législation actuelle apparaît-elle à ce point inopérante ou insuffisante pour que sa modification Et l'atteinte au droit de grève est-elle adaptée aux objectifs que l'on vise ? Surtout, ces objectifs autorisent-ils à restreindre un droit constitutionnel, chèrement acquis à grand renfort de luttes sociales Ce droit fondamental, au cours de notre histoire, aura permis aux salariés de notre pays d'obtenir des avancées ou de corriger des réformes qui leur étaient excessivement défavorables. L'exemple, pris au hasard, de la mobilisation massive contre la réforme des retraites en 1995 le montre bien, avec ses 5 millions de jours de grève cumulés et les 2 millions de personnes dans la rue le 12 décembre 1995 ... Issu du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, je puis par ailleurs témoigner de mobilisations ouvrières historiques, réprimées parfois dans la violence militaire et dans le sang, qui méritent tout notre respect et toute notre considération, et qui commandent la plus grande prudence chaque fois que l'on s'interroge sur leur restriction. Sur le fond du texte qui nous est soumis, j'aimerais partager avec vous plusieurs réflexions et interrogations. En premier lieu, sur un sujet aussi important, on ne peut regretter que la proposition de loi ne soit pas sous-tendue par une étude d'impact préalable. Je n'ai pas parlé de référendum ... Une telle étude aurait permis, sans nul doute, d'évaluer ses avantages, mais aussi ses inconvénients, tout autant que sa faisabilité. En second lieu, je reste convaincu qu'il ne nous faut pas légiférer à l'excès sur un sujet de cet ordre. Au contraire, nous devons faire confiance à l'intelligence collective, ainsi qu'à l'arsenal des règles existant d'ores et déjà. On nous dit que ces règles seraient inefficaces, car elles ne permettraient pas d'assurer un service minimum en cas de grève massive. Le taux de 90 % a même été avancé par certains ... Je suis de ceux qui pensent qu'une mobilisation d'une telle ampleur ne doit pas nous amener à imaginer quelle restriction apporter au droit de grève, mais plutôt à réfléchir au bien-fondé d'une réforme qui soulève une telle unanimité contre elle. Vous l'aurez compris, j'estime que la restriction proposée est disproportionnée. La référence au tiers des dessertes quotidiennes aux heures dites « de pointe » l'était tout autant, mais j'avoue ne pas forcément être rassuré par le texte issu de la commission. Et M. le secrétaire d'État a parlé de 50 La référence au tiers n'est plus présente. Le renvoi à l'évaluation par l'autorité organisatrice du niveau de desserte suffisant peut induire, certes, une exigence moindre, mais aussi, pourquoi pas, plus importante. En outre, la notion de période de pointe apparaît elle-même complexe à définir et sujette à interprétation, ce qui pourrait laisser présager d'importantes difficultés pratiques dans sa mise en oeuvre. Au-delà, la proposition de loi autorise la réquisition d'agents des entreprises de transport, au motif que le service minimum, tel qu'il existe aujourd'hui, serait inefficace. La logique du texte est donc bien- pardonnez-moi l'expression -une casse du droit de grève, à laquelle je ne peux souscrire. Je me permets de rappeler que la réquisition est une décision forte, privant les salariés de l'exercice de leur droit de grève et les exposant à des sanctions disciplinaires en cas de refus. Il faut donc l'autoriser avec la plus grande mesure S'engager sur la voie d'un tel durcissement des restrictions au droit de grève pourrait ouvrir la porte à d'autres velléités ... Avec, il y a lieu de le craindre, la mise en débat d'autres propositions de lois limitant le droit de grève dans d'autres secteurs affectant les déplacements de nos concitoyens, comme le transport routier, les raffineries ou encore les ports. Je comprends l'exaspération des Franciliens et de tous nos concitoyens qui ont subi les inconvénients de cette grève d'une amplitude et d'une durée rares dans notre pays, mais à qui la faute ? Y répondre par la restriction du droit de grève emporte, à terme, le risque de vider ce droit Si faire grève n'entraîne plus aucune gêne, la grève ne sera plus un moyen de pression et condamnera, au bout du compte, tout rapport de forces entre opposants et défenseurs d'une réforme. Et que dire sur l'amende forfaitaire possiblement infligée à l'entreprise défaillante ? Une nouvelle fois, les auteurs du texte se positionnent du côté de la sanction dans un champ qui relève, selon moi, prioritairement et principalement de la négociation. Il vous sera aisé de comprendre que, pour toutes ces raisons, je ne suis pas non plus favorable à l'extension du service minimum à d'autres secteurs, comme le prévoit le texte pour les transports maritime ou aérien. Les articles 9 et 10 nouveaux, ajoutés par la commission saisie au fond, introduisent la caducité du préavis de grève et la possibilité d'imposer une grève sur toute la durée du service. Ils n'emportent pas non plus mon adhésion, dès lors qu'ils reflètent cet esprit de contrainte et de restriction que j'ai pu dénoncer auparavant. Enfin, même si cela peut apparaître anecdotique à l'échelle du texte, l'article 6, consacré à l'amélioration des modalités de dédommagement des usagers, mérite qu'on le soutienne. Pour conclure, mes chers collègues, je ne suis pas opposé au service minimum, ou encore à l'encadrement du droit de grève, mais j'estime que les mesures inscrites dans cette proposition de loi ne sont ni opportunes ni justifiées.

nous nous accorderons sur un point : les sujets qui nous réunissent aujourd'hui sont complexes. J'emploie le pluriel à dessein : il traduit la réalité des enjeux que soulève cette proposition de loi et qui doivent, tous, être considérés par le législateur que nous sommes. d'abord, un constat, que nous partageons avec les auteurs de la proposition de loi. La grève qui a frappé les services publics de transport à la suite de la mobilisation du 5 décembre dernier a pesé sur notre pays. Elle a pu, en particulier, léser les plus modestes, ceux qui ne disposent pas de moyen de transport alternatif, ceux dont l'emploi ne permet pas toujours d'avoir recours au télétravail. Dans le même temps, il y a le droit. Et, plus spécifiquement, le droit de grève. Celui-ci Celui-ci s'exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent » et qui doivent, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, le concilier avec d'autres droits fondamentaux, tels que la continuité du service public, cela dans une logique de proportionnalité. C'est justement dans ce cadre que le législateur est intervenu en 2007, avec la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres. Voilà d'où part la présente proposition de loi, mes chers collègues. D'une réalité complexe, donc, à laquelle nous devons appliquer, autant que faire se peut, une approche nuancée,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 ainsi que son évolution après examen en commission, laisse à penser qu'il s'agit là d'une « réponse » plutôt que d'une « solution », pour poursuivre avec la terminologie précitée. Initialement, la proposition de loi prévoyait ainsi la définition légale d'un service minimum de transport terrestre, maritime et aérien de personnes, correspondant à un tiers du service normal. Était également prévue la réquisition des personnels non grévistes par les entreprises de transport en cas d'impossibilité d'assurer ce niveau de service. Le dispositif a nécessairement été assoupli lors de l'examen en commission. En effet, il n'apparaissait pas proportionné et présentait donc un risque sur le plan de sa constitutionnalité. Par ailleurs, il privait de leur faculté d'appréciation les AOT, qui, dans de nombreux cas, relèvent de l'échelon territorial. Or, nous le savons bien au sein de cette assemblée, cette faculté d'appréciation qu'ont les AOT est pertinente, car elle est fondée sur une connaissance du territoire et des besoins de la population. Elle apparaît par là même comme une condition nécessaire au caractère proportionné des limitations du droit de grève. Finalement, après assouplissements, le texte que nous examinons aujourd'hui dispose, comme c'est actuellement prévu par le code des transports, qu'il revient à chaque AOT de déterminer le niveau de service minimum. Autres assouplissements : la suppression de l'amende prononcée par l'AOT à l'encontre des entreprises de transport, ou encore le rétablissement de la définition contractuelle des modalités pratiques de remboursement. Enfin, la faculté de réquisition est conservée, mais ne peut intervenir qu'après injonction de l'AOT, qui ne peut elle-même être prononcée qu'après un délai de carence de trois jours. L'évolution importante dont a fait l'objet la présente proposition de loi témoigne d'un déficit de recul. Or le temps de la réflexion, cher à la Haute Assemblée, est indispensable à l'analyse d'une situation complexe ayant des implications juridiques et pratiques non négligeables. D'autant que le niveau de service minimum défini par l'AOT serait désormais au fondement d'une faculté de réquisition du personnel, ce qui implique une attention particulière au regard du droit constitutionnel. L'extension, en commission, de l'obligation d'exercer le droit de grève pendant toute la durée du service peut également poser question, eu égard à la différence de situation des salariés des entreprises de transport et des fonctionnaires territoriaux. Cette mesure aurait dû impliquer, en tout état de cause, une étude de son impact juridique. Nous pourrons probablement trouver un point d'accord sur la nécessité de mener une réflexion quant au bilan de la grève qu'a connue notre pays ces dernières semaines. une telle réflexion ne peut qu'être approfondie et s'inscrire dans un temps réfléchi et apaisé. Le droit en vigueur offre à ce titre un levier, en prévoyant que les entreprises de transport établissent un bilan annuel, détaillé et rendu public des incidences financières de l'exécution des plans de transport. Il est même précisé qu'elles doivent dresser la liste des investissements nécessaires à l'amélioration de la mise en oeuvre de ces plans. Aussi, mes chers collègues, force est de constater qu'il n'y a pas de vide juridique en matière de continuité du service public des transports. La loi de 2007 mentionnée précédemment permet d'organiser le service en amont, pendant et en aval des perturbations prévisibles du trafic, dont la grève est une composante. Est notamment prévue la définition d'un plan de transport adapté aux dessertes prioritaires, ainsi qu'un accord collectif de prévisibilité du service applicable. Notons que cet accord va jusqu'à organiser la réaffectation des personnels non grévistes, en fonction des besoins du service concerné. Soulignons également, à titre d'exemple particulièrement significatif, l'existence du contrat entre la RATP et Île-de-France Mobilités, qui prévoit la mise en oeuvre d'un service minimum équivalant à 50 % du service normal. Ainsi, avant d'entreprendre toute démarche législative, réfléchissons attentivement à la mise en oeuvre du droit en vigueur, telle que les récents mouvements sociaux Plus spécifiquement, axons cette réflexion sur les négociations conventionnelles et le dialogue social. Cette dimension sociale constitue en effet un véritable « hors champ » du texte initial, alors même qu'elle est centrale dans la loi de 2007 et qu'elle se trouve au fondement de la mise en oeuvre du service minimum. Il est difficilement envisageable de changer de paradigme sans étudier l'impact que cela aurait ou sans même consulter les personnes morales aujourd'hui compétentes. Pour conclure, mes chers collègues, ne dressons pas de vaines oppositions entre ceux qui, soutenant la proposition de loi, seraient pour l'ordre et du côté des usagers, et ceux qui, exprimant des réserves sur le texte, seraient en faveur du blocage du pays et de la dégradation de la situation. la vocation de la loi est d'être non pas performative, mais bien normative. Dire qu'une proposition de loi « répond aux besoins essentiels du pays en cas de grève » ne revient pas à répondre de manière effective aux besoins essentiels du pays en cas de grève. En témoignent les évolutions de la proposition de loi : lors de son examen en commission, le dispositif s'est justement révélé peu proportionné aux besoins pourtant mentionnés dans son intitulé. mentionnés dans son intitulé. De même, ne pas voter un texte ne revient pas nécessairement à s'opposer à son objet. L'enjeu est dans le contenu normatif. Ainsi, une approche nuancée n'est pas réductible à une position tiède, fébrile ou circonstanciée politiquement. En tant que législateur, nous devons être à la hauteur du réel et de sa complexité, ne pas confondre précipitation et réactivité. Il faut conclure, mon cher collègue. Si nous partageons les préoccupations des auteurs du texte, nous ne partageons pas les réponses que celui-ci prévoit. C'est pourquoi le groupe La République En Marche s'abstiendra.

Deuxièmement, notre groupe affirme avec conviction- il l'a prouvé à maintes reprises -l'importance qu'il accorde à tous les corps intermédiaires et au dialogue social social : si la grève permet d'appuyer des revendications professionnelles, c'est avant tout le dialogue qui résout 60 % et plus des conflits sociaux dans les entreprises et les services publics. Troisièmement, les législateurs que nous sommes doivent tout à la fois- cela a été réaffirmé par un certain nombre d'orateurs -défendre les intérêts des professionnels et également sauvegarder l'intérêt général auquel la grève peut parfois porter atteinte. Nous ne devons pas le nier, car cela revient parfois à oublier les plus faibles d'entre nous.

ans se sont écoulés depuis. Entre-temps, le climat social a évolué. S'est-il durci ou pas ? Chacun en jugera ! En tout cas, les modes d'expression ont changé. Il faut le dire, certains syndicats ont su faire preuve de beaucoup d'imagination pour s'adapter à cette loi. Les grèves de cinquante-neuf minutes, qui ont été évoquées, les grèves dites « longues » ou « illimitées » n'en sont que des exemples ; j'y reviendrai. Je réaffirme donc avec force et conviction que ce texte de loi est nécessaire et attendu, et qu'il ne contrevient en aucune façon au droit de grève, qui, en France, a valeur constitutionnelle. Par ailleurs, ce texte de loi répond à des enjeux de société fondamentaux, qui visent certes à éviter les prises d'otages de nos concitoyens, mais également à donner crédit aux actions publiques de transition écologique, qui poussent à développer les transports publics en assurant

perdurent en l'absence de grévistes, privant d'effet les dispositions prévues par la loi du 21 août 2007 en matière de grève. Je pense aussi aux arrêts de travail de très courte durée, qui perturbent le service et entraînent une désorganisation complète des services de transport. Je pense instaurer des mouvements de grève discontinus ingérables. Je pense enfin aux déclarations de salariés quant à leur arrêt de travail ne permettant pas d'organiser efficacement les services. L'ensemble de ces pratiques porte un préjudice considérable aux voyageurs, aux autorités organisatrices et aux entreprises de transport public de voyageurs, qui ne peuvent prévenir utilement les clients ... Les usagers ! ... en cas de perturbations de trafic. Je remercie donc Mme le rapporteur d'avoir intégré à ce texte des amendements visant à permettre à l'entreprise d'imposer au salarié gréviste d'exercer son droit durant toute la période de son service et à empêcher le recours répété à des grèves courtes ou de plusieurs décennies. En conséquence de quoi, je vous invite, sans contrevenir, monsieur le secrétaire d'État, à la mission que vous venez de nous proposer, à voter ce texte de loi, dans l'intérêt des usagers et des transports publics.

si les mouvements de grève en France sont vus à l'étranger comme un sport national, la présente proposition de loi rappelle, à juste titre, que ce droit de valeur constitutionnelle ne peut supplanter celui qui tend à assurer la continuité du service public. Je salue ainsi ce texte, qui apporte des réponses concrètes face aux récents abus du droit de grève, de tels abus posant la question de l'encadrement de ce droit, et ce pour deux principales raisons. Dans un premier temps, nous ne devons pas oublier que les difficultés quotidiennes qu'ont connues nos concitoyens ont tout ont tout d'abord affecté les plus précaires d'entre eux. Cette situation, conduisant à une véritable « galère » de travailleurs qui sont tributaires des transports publics et se retrouvent sans aucune autre solution, se traduit également sur la fiche de paie et peut avoir des conséquences dévastatrices. Il était donc indispensable de compléter la loi du 21 août 2007, afin d'assurer un véritable service minimum qui puisse lutter contre les abus du droit de grève. au manque de solutions de mobilité, de tels abus sont vécus comme une source d'inégalités et d'injustice entre les citoyens, et de fractures entre les territoires. C'est le sentiment d'une assignation à résidence pour une population sans solution Ainsi, la proposition de loi permettrait des améliorations réelles, en introduisant une exigence de service garanti en cas de grève et en luttant contre les grèves de courte durée, qui désorganisent de manière excessive le service public de transport. De même, en permettant à chaque autorité organisatrice de transport de définir le niveau de service minimal nécessaire à la couverture des besoins de la population, les apports de la commission des affaires sociales ouvrent la voie à une différenciation bienvenue, qui préfigure les débats à venir au sein de cet hémicycle. il se révèle que les abus que je dénonçais précédemment vont également à rebours des efforts engagés afin de répondre à l'urgence climatique. Tandis que la priorité doit être de transférer les passagers de la route vers le rail pour réduire les émissions polluantes, les grèves à répétition font rebasculer une partie du trafic ferroviaire sur la route. C'est un contresens

De même, en provoquant des pertes considérables, dépassant le milliard d'euros, pour un opérateur déjà endetté à hauteur de près de 55 milliards d'euros, les grèves mettent à mal les indispensables efforts d'investissements sur le rail. De tels efforts sont pourtant essentiels pour développer le fret et acter le développement de réseaux ferrés transeuropéens, mais également participer à la desserte fine de nos territoires dépendants de la voiture. Vous avez tout cassé ! Pour toutes ces raisons de justice sociale, d'urgence climatique et d'équilibre entre deux droits étroitement liés, le groupe Union Centriste votera en faveur d'une telle proposition de loi. Bravo ! La parole

L'élue de Paris et l'usagère des transports que je suis est en colère de constater le chaos auquel les Parisiens ont dû faire face depuis plusieurs mois. Ces Parisiennes et ces Parisiens auxquels la bien-pensance explique, depuis des années, que la genèse de tous les maux de la terre se trouve dans leur pot d'échappement et que la réduction de leur empreinte carbone commence par l'utilisation des transports en commun, que le développement du commerce en ligne conduira inévitablement à la mort de leur boutique de quartier s'ils ne font pas l'effort conscient d'acheter physiquement les produits qu'ils consomment, que le bien-être de leurs enfants repose sur une routine stable et équilibrée ! Je parle au nom des dizaines de milliers de Parisiens qui, pendant un mois et demi, ont été contraints de marcher en moyenne dix kilomètres par jour pour maintenir leur activité professionnelle, de ceux qui ont développé tous les symptômes physiques et psychologiques du fameux burn-out, dont le Gouvernement entendait entendait faire une priorité de santé publique, des enfants dont le temps de sommeil a été bouleversé parce qu'il fallait une heure de transport de plus par jour. Eh oui ! Je parle aussi au nom des neuf commerces sur dix qui ont déploré une baisse de fréquentation et de leur chiffre d'affaires- jusqu'à 60 % pour certains,

mêmes Français qui ont subi de plein fouet le mouvement des « gilets jaunes » l'an dernier. Ils n'acceptent plus que la première région économique d'Europe, qui rassemble un tissu entrepreneurial parmi les plus denses au monde avec 1,055 million de TPE, PME, d'ETI et de grands groupes, et qui produit 31 % du PIB du pays, puisse être paralysée par un mouvement de grève, aussi légitime soit-il ! Ils n'acceptent plus non plus que l'État, comme la Ville de Paris, soit contraint de dédommager ces entreprises au moyen de de la recette de leurs prélèvements obligatoires. de leur liberté et de leur droit de se déplacer ? Personne dans cet hémicycle ne remet en question l'intégrité du droit de grève, tel qu'il est garanti par la Constitution. Si

des transports. Pascale Gruny l'explicite parfaitement dans son rapport : « Lorsqu'une activité de transport relève d'un service public, le principe de valeur constitutionnelle de continuité du service public justifie en lui-même une intervention des pouvoirs publics ». Les articles de cette proposition de loi se concentrent sur des situations de grève portant directement atteinte à la continuité du service public, voire au principe même de continuité territoriale en ce qui concerne la desserte des îles françaises. Avec la région d'Île-de-France, ces dernières sont les grandes perdantes des blocages à répétition, qui altèrent non seulement la possibilité d'aller et de venir des citoyens, mais également leur approvisionnement. Cela a été notamment le cas en Corse, ces trois dernières semaines, où des rayons entiers de supermarchés étaient Les dispositions relatives au transport aérien prévues aux articles 8 et 9 tendent à répondre aux mêmes problématiques et affectent notamment l'accès aux soins de nombre de nos compatriotes, contraints de prendre l'avion pour bénéficier de certains traitements médicaux. Enfin, les articles 5 et 6 tendent à prévenir les situations de chaos auxquelles nous assistons en cas d'opérations coup de poing et de blocages intempestifs. Une communication entre l'entreprise de transport et l'autorité organisatrice du mouvement de grève est indispensable, afin d'assurer une information fiable des usagers. De même, tout titre de transport non utilisé doit être remboursé le moyen de paiement qui a été utilisé, et non par un échange ou un avoir. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement de Valérie Pécresse, présidente de la région d'Île-de-France, afin de s'assurer que chaque usager est remboursé de son pass Navigo pour le mois de décembre. Dans cet hémicycle où nous examinons régulièrement des dispositions éminemment techniques, pour ne pas dire parfois technocratiques, je le dis clairement : il n'y a rien de plus concret, me semble-t-il, que d'assurer aux Français la possibilité de se déplacer. Je remercie donc Bruno Retailleau d'être à l'initiative de ce texte. La parole

Respectueux de la Constitution qui consacre la grève comme un droit, nous ne pensons pas que cette dernière puisse être définie comme une perturbation prévisible- article 2 -ni qu'elle puisse être déclarée caduque- article 9 -ou empêchée- article 10. Au reste, ce dernier article ajouté en commission m'interroge vraiment du point de vue constitutionnel, puisqu'il vise à empêcher le recours à des grèves de courte durée.

Éviter au maximum les perturbations, notamment dans la durée, pour les usagers passe selon nous, tout d'abord, par une nouvelle approche et un véritable dialogue social. L'article 3 ne ferait en tout état de cause que jeter de l'huile sur le feu, comme l'ensemble de ce texte, qui a pour seule vocation de poser un marqueur politique. Avec l'article 1, vous souhaitez étendre le champ d'application de la loi de 2007, dont nous estimons qu'il est bien suffisant. Quant aux procédures d'information et de remboursement des voyageurs- articles 5, 6 et 7 -, si elles sont souhaitables, elles ne peuvent servir de faire-valoir à la déstabilisation totale du droit de grève

Nous ne tomberons pas dans le piège que vous nous tendez de la division entre les travailleurs ! Enfin, ce n'est pas parce que votre texte est presque exclusivement centré sur le ferroviaire que nous laisserons passer des atteintes au droit de grève dans le secteur aérien, été largement remodelé et réduit à pas grand-chose par la commission, qui a bien vu la fragilité juridique du dispositif : à défaut d'une étude d'impact, je rappelle à mes collègues que les lignes soumises à des obligations de service public ne sont qu'une dizaine en France. preuve que vous n'avez pas cherché à répondre concrètement et complètement aux problématiques des usagers des transports. « Assurer l'effectivité du droit au transport », dites-vous ?

remercie les grévistes, qui ont supporté quarante-cinq jours de grève illimitée, pas par plaisir ni par sadisme. Et la loi El Khomri ? Ils ont fait grève par délégation pour tous les Français qui ne veulent pas de cette mauvaise réforme des retraites.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je suis un ardent défenseur d'un principe fondamental, qui, à mon sens, devrait constituer le ciment de notre société et la valeur cardinale du vivre ensemble, la liberté des uns doit s'arrêter là où commence celle des autres. Très bien ! Certes, nous avons la chance, dans notre pays, de disposer de droits fondamentaux inscrits dans le marbre de notre Constitution. néanmoins de constater, à la lumière des blocages observés ces derniers mois, que ces droits peuvent entrer en quelque sorte dans une concurrence insoluble si on ne les réglemente pas. Ainsi, le droit de grève, appliqué au secteur des transports, entre en conflit avec la liberté des Français d'aller et de venir à leur guise, de poursuivre leurs activités, de quelque nature qu'elles soient, et évidemment, en premier lieu, de se rendre à leur travail. Rappelons que, pendant les grèves du mois de décembre dernier, certains de nos concitoyens ont été contraints d'interrompre leur activité professionnelle, de prendre des congés- payés ou non -ou de renoncer à des déplacements stratégiques. Les conséquences financières ont été importantes pour beaucoup, notamment les plus fragiles. Cela a aussi eu un impact sur la croissance de notre pays, qui n'a franchement pas besoin de handicap supplémentaire dans le contexte actuel. La présidente de ma très belle région des Pays de la Loire, Christelle Morançais, a pleinement conscience de cet enjeu et proposait, il y a tout juste deux mois, une obligation de circulation pour au moins un tiers des trains. Elle suggérait même une obligation totale la veille des vacances scolaires, à l'instar de ce se pratique déjà depuis plus de vingt ans en Italie. Je salue donc l'initiative courageuse de Bruno Retailleau et le travail méticuleux de Mme la rapporteure Pascale Gruny pour aller dans ce sens et produire cette proposition de loi, qui s'attaque à un sujet délicat, que d'aucuns voudraient ériger en tabou absolu. absolu. C'est un texte mesuré, qui prend en compte les réalités exposées précédemment et qui, bien évidemment, n'est pas contraire à notre Constitution. Oui, le droit de grève est un droit fondamental, mais il peut être réglementé. D'ailleurs, cela s'est déjà fait dans notre pays, par exemple dans l'enseignement primaire. Par les décisions qu'il a rendues, le Conseil constitutionnel a renforcé l'habilitation du législateur à fixer des limites au droit de grève, à concilier la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut porter atteinte. C'est la traduction opérationnelle du septième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. D'un point de vue politique, je veux souligner la position paradoxale de quelques-uns de nos collègues. En effet, on ne peut pas clamer haut et fort son attachement au service public, sa conviction qu'il est indispensable au bon fonctionnement de notre activité humaine, et, en même temps, si j'ose dire, nier la nécessité de sa continuité, contester son utilité à chaque instant ! Si la grève apporte évidemment son lot d'inconforts, voire de nuisances, elle ne peut pas, elle ne doit pas pénaliser l'ensemble d'une population ayant à subir la force de paralysie d'une minorité, quels que soient ses motifs de protestation. On peut même aller plus loin, sans vouloir donner de leçons aux leaders syndicalistes qui, de toute façon, n'entendent généralement pas grand-chose : il y a fort à parier qu'une grève qui n'entraverait pas les droits des usagers aurait tendance à être plus populaire et mieux acceptée. Elle susciterait même davantage d'adhésion. Enfin, comment de ne pas admettre unanimement que les blocages dans le secteur du transport de passagers vont totalement à l'encontre des intentions de la transition souhaitée dans le domaine des mobilités ? Comment ne pas comprendre que, pour changer durablement les comportements, pour créer des habitudes, il est indispensable de pouvoir faire confiance à ce service public censé assumer les orientations inscrites par exemple dans la dernière loi d'orientation des mobilités ? Pour faire consensus sur ces objectifs de bon sens, je vous appelle à voter sans réserve cette proposition de loi ! La discussion

pour présenter l'amendement n° 24. Le présent article prévoit l'application du service garanti aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises, ce qui recouvre non seulement les îles métropolitaines, mais aussi les îles d'outre-mer dans la mesure où le code des transports y est applicable. La commission a complété ces dispositions en étendant aux services de desserte maritime des îles les dispositions relatives au dialogue social, à la prévention des conflits collectifs et à l'exercice du droit de grève qui sont applicables aux services de transport ferroviaire issu de la loi de 2007. C'est donc tout un processus nouveau autour de l'usage du droit de grève par le système de déclaration individuelle, de prévention des conflits, de durée du préavis pour l'instauration d'une sorte de « préavis du préavis » et d'organisation particulière de service. Autant de règles à nos yeux profondément attentatoires au droit de grève, et ce sans aucune étude d'impact et sans avis du Conseil d'État. Cela ne nous paraît absolument pas sérieux. Comment engager de telle restriction d'un droit fondamental sans même prendre la peine d'entendre les acteurs de ce secteur d'activité et les partenaires sociaux ?

l'avait rejeté pour un double motif : la faible conflictualité au sein des transports maritimes et la liberté des collectivités territoriales dans le cadre des contrats de délégation de service public, qui, pour la plupart, contiennent déjà des dispositifs d'alarme sociale pour prévenir les conflits. Même Nicolas Sarkozy, qui a eu l'initiative du texte relatif au service minimum, en 2007, avait renoncé à y inclure les transports maritimes pour les mêmes motifs. les mêmes motifs. Puisque tout le monde s'accorde sur la nécessité de ne pas étendre ces mesures aux transports maritimes, nous demandons le rejet de cette disposition purement démagogique.

... Le socle de cette proposition de loi, c'est l'instauration d'un service dit « garanti », et non plus « minimum », par la possibilité de réquisitionner les salariés nécessaires à l'accomplissement des besoins définis comme essentiels par l'autorité organisatrice.

est d'ailleurs incroyable de voir ceux-là mêmes qui ont ouvert la SNCF et la RATP à la concurrence pleurer, aujourd'hui, la continuité du service public. C'est même un comble

Cette proposition de loi constitue une véritable provocation sociale, dans un contexte déjà particulièrement tendu, à cause de la volonté inébranlable de faire passer en force le projet de loi portant Toute la communication institutionnelle, relayée par les médias, tend à faire passer les grévistes pour des fauteurs de troubles irresponsables, guidés par la seule volonté de défendre leurs acquis, sans visée collective. C'est évidemment faux : les grévistes, notamment dans les transports- qui paient le plus lourd tribut à la lutte -, se battent pour tous, y compris pour ceux qui ne font pas grève aujourd'hui. Ils sont les « premiers de cordée » de la forte contestation sociale que connaît notre pays. En exerçant leurs droits,

D'ailleurs, une forte complicité se fait jour entre le Gouvernement et les directions d'entreprise pour casser les droits collectifs des travailleurs, que ce soit en mettant fin au statut, par de précédentes réformes, comme le pacte ferroviaire, ou en brisant les grèves, y compris en accordant des primes

grève les agents du service public de transport en organisant les conditions de leur réquisition, c'est nous condamner collectivement à renoncer à tout grand progrès social. Nous demandons donc le retrait de cette proposition de loi, qui- nous le répétons -est une provocation, surtout dans le moment social que nous sommes en train de vivre. La parole est à Mme Laurence Cohen,

pour financer les services publics, pour que, enfin, ce ne soit plus la galère quotidienne dans les transports. Vous le savez comme moi, les grèves constituent une part infime des dysfonctionnements.

Il est totalement démagogique de pointer du doigt les grévistes pour leur imputer tous les maux de la dégradation du service public. Comment ignorer que ces agents se mobilisent, justement, pour la sauvegarde de leur outil de travail,

celui de l'utilité des agents publics et des services publics. Il faut transmettre le message à tous ceux qui, hypnotisés par le dogme de la réduction de la dette, veulent supprimer des emplois, que ce soit parmi les fonctionnaires de l'État ou dans les entreprises publiques, notamment à la SNCF.

Certains ont même affirmé que les luttes, les grèves et les occupations d'usines auraient permis le progrès social. Regardez et écoutez le peuple qui est dans la rue aujourd'hui C'est un peuple qui se bat, car il souffre. Toutes ces personnes expriment leur mal de vivre, refusent la baisse du pouvoir d'achat. Ils défendent leur travail, demandent des augmentations de salaire, une meilleure retraite. Ils rejettent en bloc les lois qui s'attaquent à leurs acquis sociaux, comme le droit du travail ou le droit à la retraite. Maintenant, vous voulez même les empêcher de s'exprimer, en encadrant par ce texte un service minimum pour que le pays ne soit plus bloqué. Allez-y, chers collègues,

! Lesquelles ? Réfléchissez-y, et vous verrez que notre demande de suppression de ce texte est primordiale

est le dernier recours. Quand les électriciens se mettent en grève, il n'y a pas de courant. Quand les cheminots et les traminots se mettent en grève, il n'y a pas de transport. Quand les professeurs se mettent en grève, il n'y a pas de cours. C'est ainsi, mais ne croyez pas que c'est par plaisir qu'ils le font.

une mission de continuité du service public, et admettre l'idée qu'il puisse ne pas y avoir de service public des transports dans le pays pendant des semaines. Cela revient à nier la mission de service public et de continuité du service public de ces entreprises. C'est vrai ! Il faut donc trouver un équilibre entre

sans avoir ensuite la responsabilité de mettre en place le service minimum. Oui, il faut un équilibre entre le droit de grève et la continuité du service public. Eh oui, cela dépend entièrement des régions autorités organisatrices La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote.

de pénalités financières. Nous ne savons pas comment elles pourront faire respecter cette obligation : j'espère qu'elles ne pourront pas faire appel à la force publique, qui reste heureusement encore un pouvoir régalien. De même, nous ne connaissons pas les conséquences

que l'article n'est pas satisfaisant. C'est bien pour cela que nous souhaitons le supprimer ! Par ailleurs, dans votre exposé liminaire, vous avez livré un chiffre, qui est extrêmement intéressant, dans le grave conflit

Je voudrais que l'on soit précis sur ce que l'on vote. J'ai entendu dire tout à l'heure que le texte ne faisait jamais qu'élargir ce qui existait déjà. En l'état actuel du droit, aucune entreprise privée ne peut procéder à la réquisition des salariés, c'est de jurisprudence constante. Or le service public des transports n'est pas uniquement assuré par des entreprises publiques. Si l'on en croit d'autres débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle précédemment, il existe une forte volonté

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement constate que le Conseil d'État s'est fondé à plusieurs reprises et de façon assez constante sur la durée du mouvement pour juger de la validité d'une réquisition et, dès lors, supprimer tout délai qui serait de nature à fragiliser

d'abord, vous décrivez un paysage social assez monolithique, qui ne ressemble pas à ce que j'ai pu vivre au contact des syndicats. Vous décrivez des syndicats qui seraient unanimement contre la réforme des retraites. J'ai eu affaire à des syndicats qui, pour partie, pratiquaient ce qu'ils ont qualifié eux-mêmes de « réformisme combatif » : sans être

dans le respect du droit. Cela n'implique pas, par exemple, un droit de retrait abusif ou des pressions sur des collègues. C'est faux ! Je vous rappelle que des procédures disciplinaires sont en cours, qui sont particulièrement graves.

permet déjà au préfet de réquisitionner tout service ou tout bien et de requérir toute personne pour assurer l'ordre public. Or ces dispositions

effet, c'est bien d'une nouvelle attaque contre le droit de grève qu'il s'agit. En outre, on stigmatise une fois de plus les salariés des transports publics, en particulier les cheminots et les chauffeurs de bus, dont les conditions de travail sont particulièrement pénibles, car ils travaillent régulièrement le samedi et le dimanche, les soirs ou les nuits. que les chauffeurs de bus en Île-de-France sont régulièrement confrontés à des incivilités et à des violences. On comprend donc qu'ils puissent être attachés à leur statut et à leur régime spécial de retraites, qui peuvent être vus comme des compensations légitimes eu égard à la pénibilité de leur métier. Pourquoi, selon vous, la RATP a-t-elle autant de mal à recruter des chauffeurs de bus, si ce n'est en raison de la pénibilité de ce métier ? Pensez-vous qu'il soit opportun d'examiner une telle proposition de loi après un conflit aussi dur,

Votre proposition de loi relève du pur opportunisme politique. Nous nous opposons à cette nouvelle attaque contre le droit de grève. Ce n'est pas sérieux ! Il n'y a pas que les salariés des transports publics qui se sont mis en grève de nombreux autres secteurs d'activité sont aujourd'hui touchés par des mouvements de grève. Ces salariés sont eux aussi inquiets pour l'avenir de leur régime de retraite, pour eux et pour leurs enfants. Si vous stigmatisez les cheminots et les chauffeurs de bus, c'est parce que les désagréments qu'ils causent aux usagers sont sans doute plus visibles que dans d'autres secteurs et que vous jouez sur l'exaspération de certains de nos concitoyens. Ce n'est pas à la hauteur de la situation actuelle et de la grogne sociale qui monte, alors que de nombreux salariés, dans de multiples secteurs d'activité, se sont mis en grève ces derniers mois. Ils sont inquiets, alors que les inégalités sociales ne cessent de croître et que les mesures du Gouvernement participent d'un mouvement de régression

de bus délégataire d'une communauté d'agglomération, par exemple, fera-t-elle pour informer l'agglomération en question de l'avancée des négociations entre les syndicats

l'avis du Gouvernement ? Dans le droit fil de ce que vient de dire Mme la rapporteure, je rappelle que le code des transports prévoit déjà des plans de transport à l'article L. 1222-4, lesquels définissent des niveaux de service minimum. Par ailleurs, si ces plans de transport ne sont pas respectés, l'article L. 1222-11 prévoit

Ces comités associent aujourd'hui les représentants des usagers, des personnes handicapées et des élus locaux. Ils sont utiles pour améliorer le service public des transports, notamment ferroviaires, pour garantir une réelle présence territoriale et pour lutter contre les velléités de rétraction du réseau sur les axes rentables

la qualité de service, la performance énergétique et écologique et la définition des caractéristiques des matériels affectés à la réalisation des services ». Mes chers collègues, nous ne pouvons accepter que ces comités deviennent des outils de restriction du droit de grève

de transport aérien placées sous obligations de service public. Je rappelle que la loi sur le service minimum dans les transports terrestres de voyageurs ne s'applique pas au secteur aérien, et ce pour une raison évidente : la plupart des lignes aériennes ont été libéralisées et n'assurent

Enfin, mes chers collègues, comment ne pas relever votre manque de cohérence politique ? Vous donnez compétence au ministre chargé de l'aviation civile d'imposer, sur proposition des collectivités territoriales, une obligation de service public sur certaines lignes

ce faisant d'empêcher le recours répété à des grèves de courte durée, qui constitue pourtant l'une des modalités du droit de grève. Une telle restriction porte une fois de plus une atteinte manifestement disproportionnée au droit de grève. Aujourd'hui, la réglementation autorise les agents à faire grève sur une période d'une heure ou sur une période de quatre heures, précisément cinquante-neuf minutes pour le premier cas et trois heures Ces dispositions peuvent s'opérer uniquement à la prise de service de l'agent, et pas en cours de journée de travail. Cela permet de ne pas trop gêner le service public

le service. Le décompte de salaire s'effectuant sur la période en heures de grève réalisées, et non sur une journée de travail complète, cette modalité d'exercice du droit de grève est moins lourde financièrement pour ceux qui y recourent. En tout état de cause, en rendant l'exercice du droit de grève plus difficile, une telle atteinte à un droit constitutionnellement garanti est inacceptable.

part, je ne perçois pas cette proposition de loi comme restreignant l'exercice du droit de grève. Je crois au contraire qu'elle s'inscrit dans un esprit d'équilibre. Nous sommes face à une situation qui est aujourd'hui

à l'hémicycle, n'est absolument pas satisfaisant. Les entreprises privées n'auront pas la capacité d'exercer ce transfert et cette cette réquisition, sinon en faisant appel à la force publique. J'ai apprécié les interventions de ma collègue Michèle Vullien, qui a rappelé que le recours à la force publique devait rester un pouvoir régalien de l'État ; sinon, où allons-nous ?